L'Ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi tendante à renforcer la culture citoyenne présentée par M. Henri Cabanel et plusieurs de ses collègues. du groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Dans la discussion générale, la parole est à monsieur Henri Cabanel, auteur de la proposition de loi.

Monsieur le Président, excusez-moi. Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission de la Culture, Monsieur le rapporteur, Mes chers collègues, savez-vous ce qu'est la citoyenneté ? 28 % des 628 jeunes du lycée Henri IV de Béziers et 218 du lycée Pro Mermos, qui ont répondu à une enquête que j'ai initiée avec leur enseignant, M. Fonteret et Mme Kierdermans, ont répondu oui. un chiffre qui ferait frémir les rédacteurs de la déclaration de l'homme et du citoyen. En 1789, ils affichaient ainsi leur motivation. Les représentants du peuple français, constitués en assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappel sans cesse leurs droits et leurs devoirs. afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique en soient plus respectés. Afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. Deux siècles et demi plus tard, qu'est devenu la notion « bonheur pour tous » ? Alors que la défiance des citoyens envers leurs élus et leurs institutions n'a jamais été aussi exacerbée, il me semblait utile de se poser la question et de se remettre en question. Car les différentes analyses s'accordent au moins sur les constats. En mars 2023, 75% des Français interrogés dans le cadre du dernier baromètre Sevipov disent de ne pas faire confiance au gouvernement. Nous ne sommes pas loin derrière, nous les parlementaires, avec une défiance entre 68 et 72 %. À cela s'ajoute la progression des agressions des élus, après une hausse de 32 % en 2022. À cela s'ajoute la place grandissante accordée aux réseaux sociaux. Après les élus, les journalistes subissent eux aussi une perte de confiance. Dans un sondage candar public, One point pour la Croix, 57% des Français pensent que la plupart du temps, il faut se méfier de ce que disent les médias sur les grands sujets d'actualité. Dans ce contexte de défiance, comment revenir aux valeurs communes de notre République ? Mon groupe RDSE a bien compris l'enjeu principal de ce travail. Se réunir autour des valeurs et aller vers un avenir partagé, je l'en remercie. La mission, présidée par notre collègue Stéphane Piennoir, s'est structurée autour de trois axes principaux. Mieux éduquer, encourager une citoyenneté active, repenser les pratiques démocratiques pour rapprocher les citoyens des institutions. Tout d'abord, bien éduquer. Fort du constat de défiance des citoyens, nous avons opté pour un parti pris, nous préoccupés des jeunes. Car la citoyenneté se construit, elle s'enseigne, elle s'apprend. L'éducation morale et civique a donc été le point central de notre travail. Avec un constat, les réformes successives ont entraîné une instabilité de la matière. Dans une conférence en 2018, Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d'État, indique bien que la réforme de l'MEC soit érigée au rang de priorités politiques de l'exécutif, la discipline se voit en fait attribuer des moyens limités et garde un statut très secondaire. Deux de ces avis me semblent essentiels. Le premier, développer et maintenir les liens réciproques entre les jeunes, les institutions républicaines et les organisations de la société civile. J'ai d'ailleurs initié dans mon département un projet d'intervention de binôme d'élus dans les établissements scolaires. Certains m'auront torqué, mais on le fait tous. Non, on ne le fait pas tous. Et pas de façon structurée, pas de façon encadrée. La convention consignée récemment avec Sophie Bégin, rectrice de l'Académie de Montpellier, et Frédéric Roig, président de la MF 34, énonce les enjeux. Les élus vont porter d'une même voie, auprès des jeunes scolarisés, les valeurs de la République, les droits et les devoirs. C'est plus symbolique que dans un pays où désormais les enseignants sont cible d'actes terroristes générés par l'obscurantisme. Jean-Marc Sauvé explique la refondation du pacte de citoyenneté devrait passer en premier lieu par la réaffirmation des valeurs qui sont à sa racine. La citoyenneté française s'est escrite dans une vision partagée du bien commun et de l'intérêt général. L'individualisation et l'émiétement de nos sociétés abolissent les intermédiactions et conduisent les citoyens à se replier sur des choix individuels. C'est pourquoi je suscris pleinement à sa deuxième proposition d'intégrer les jeunes en un monde à la construction des politiques publiques qui les concernent. Car la citoyenneté se construit à l'école. L'égalité des chances n'est pas la même quand on sait que seulement 10% des Français indiquent que l'orientation dans la voie professionnelle est choisie. Comment se sentir citoyen, c'est-à-dire partie prenante de la société quand on vit dans un quartier qui concentre un grand nombre de difficultés ? C'est pourquoi je travaille à ce sujet avec une trentaine de jeunes de Belieu, de Voie-en-Velin, de Paris, de Marseille, de Toulouse, grâce à la motivation de Dylan Aissy, un jeune engagé qui a créé l'association Une Voie Pour Tous. Tout au long de notre mission, nous avons évidemment auditionné des experts, mais celles dont je suis le plus fier, ce sont celles des jeunes. Car parler des jeunes sans parler aux jeunes, sans écouter les jeunes, sans se nourrir de leurs réflexions, de leurs idées, cela ne sert à rien. J'ai organisé un déplacement dans mon département dans le quartier populaire de Montpellier, la paillade. Les sénateurs ont entendu, les jeunes parlaient de leur vie, la vraie vie. L'un d'eux a dit « je me sens exclu de la République ». Comment se sentir citoyen quand on se sent exclu de la République ? Deuxième axe de notre mission, encourager une citoyenneté active. Pour faire une société, le citoyen doit se sentir acteur de son devenir. C'est dans cet esprit qu'a été créé le service civique héritier direct du service civil volontaire créé par une loi dont le projet a été déposé. Ce point est éclairant quelques semaines après les violentes émeutes des balieux de 2005. Plus récemment, la création du service national universel s'est escrite dans une démarche similaire. Et les débats conqués sur son aspect militaire ne sont que de faux arguments. L'urgence du contexte nous impose d'être unis à ce sujet contre des idées fausses. Tant le service civique que le SNU considère l'engagement des jeunes comme le socle de leur formation citoyenne. C'est pourquoi je suis favorable à les faire cohabiter. À l'heure de la montée en puissance du SNU, ce serait une erreur d'abandonner le service civique. Il faut, au contraire, le développer et le voir comme un complément. Le SNU offre les bases, le service civique les développe, les nourrit, et apporte au volontaire une expérience à la fois humaine de solidarité, mais aussi professionnelle. Dans une récente étude auprès des jeunes volontaires, Unicité, présidée par Marie Trélu-Cannes, pointe l'importance du service civique pour les jeunes décrocheurs scolaires. L'association préconise aussi de se préoccuper de la mobilité en milieu rural. Enfin, troisième axe de notre travail, repenser les pratiques démocratiques pour rapprocher les citoyens des institutions. Faire un état des lieux de notre système, c'est bien. Nous remettre en question, c'est mieux. Les Français n'ont plus confiance. Alors qu'avons-nous raté ? Les partis politiques sont à bout de souffle, mais on continue. Jusqu'à quand ? Jusqu'à quel mur ? L'abstention s'élève aujourd'hui comme le premier parti en France. Jusqu'où irons-nous sur la légitimité du suffrage universel, quand les maires des grandes villes, en 2020, ont été en moyenne élus avec 18% des inscrits ? J'aurais souhaité aller plus loin dans les préconisations, mais vous le savez, pour qu'un rapport soit voté, il faut composer. Donc j'ai composé sur la démocratie contributive qui me tient à cœur, la reconnaissance du vote blanc, le vote obligatoire, qu'il faudra bien un jour mettre en débat. Nous en sommes restés au mode de scrutin. D'autres textes, et demain la réforme institutionnelle annoncée lors du premier mandat du Président de la République, nous forcera peut-être à nous poser les bonnes questions. Cette proposition de loi est loin de poser de façon exhaustive les problèmes de la citoyenneté et des jeunes. Adoptée à l'unanimité le 7 juin 2022, le rapport de la mission d'information est assorti de 23 recommandations. Six de ces 23 recommandations supposent des modifications de dispositions législatives en vigueur concernant le MEC, la journée de défense et de citoyenneté, les EPID, la double procuration, la profession de foi électronique, le statut de l'étudiant élu. Cette PPL est donc limitée car elle n'a pour seule ambition de faire progresser quelques préconisations. Mais je me réjouis de son vote à l'unanimité en commission culture et je remercie Mon ami le rapporteur, mon collègue Bernard Fialer. Nous avons travaillé ensemble à la réécriture de certains articles qui augurent, je l'espère, très sincèrement, une avancée prouvante. C'est comme cela que je conçois le travail parlementaire en une co-construction dans le seul but d'améliorer l'existent et surtout dans le seul but de l'intérêt général. Je vous remercie. Merci, merci monsieur Cabanel. Dans la suite de la discussion générale, la parole est maintenant à monsieur Bernard Fialer, rapporteur de la Commission de la Culture. Monsieur le Président, Madame la Ministre, monsieur le Président de la Commission, monsieur l'auteur de la loi, chers collègues. Rien n'est moins naturel que la démocratie qui consiste à remplacer la violence, verbale ou physique, par des discussions, des compromis et des efforts collectifs. Ces propos de Dominic Schnapper témoignent de l'importance d'entretenir la flamme de la culture citoyenne pour que la démocratie reste vivante. Aussi, je salue les travaux de la mission d'information visant à redynamiser la culture citoyenne présidée par Stéphane Piénoir et dont Henri Cabanel était le rapporteur. Celle-ci a identifié un parcours citoyen constitué de cinq étapes clés. L'école, la journée défense et citoyenneté, vestige du service militaire, les dispositions d'insertion sociale et les élections. Parce qu'ils sont partagés par chacun, ils forment un projet collectif fondé sur des références partagées. Or aujourd'hui, chacune de ces étapes s'effrite. Par conséquent, les références partagées s'étiolent et le projet collectif se délite. Il en résulte une archipélisation de la société pour reprendre l'expression de Jérôme Fourquet. La mission d'information a cherché à identifier les mots dont souffre notre démocratie. Elle a fait 23 recommandations pour renforcer le lien entre le citoyen et les institutions. la proposition de loi de notre collègue Henri Cabanel reprend celle à portée législative. Nous en sommes tous conscients. Ce texte ne permettra pas à lui seul de réconcilier les citoyens, notamment les plus jeunes, avec la participation à la vie démocratique. Néanmoins, Il permet d'agir afin d'éduquer et de former à la citoyenneté et de repenser les pratiques démocratiques. Il y a 120 ans déjà, Ferdinand Buisson disait « Le premier devoir d'une République, c'est de faire des Républicains ». L'article premier de ce texte vise à recentrer l'enseignement moral et civique sur des objectifs concis. Je ne peux que saluer cette volonté politique. La Commission de la Culture n'a eu de cesse à chaque modification de cet article de regretter la tendance du législateur à définir dans la loi le contenu des programmes. Aujourd'hui, l'OMC souffre d'un contenu pléthorique accentué par l'absence d'heures dédiées. Cela conduit à une perte de valeur et références partagées entre l'ensemble d'une classe d'âge. En effet, par manque de temps, l'enseignant va piocher des chapitres dans le programme en fonction de ses appétances, de sa maîtrise du sujet ou ce qu'il estime intéressant pour ses élèves. Avec un enseignement dépendant des choix du professeur, pour reprendre les mots de Jean-Pierre Aubin, ancien inspecteur de l'Éducation nationale, c'est la volonté collective qui en pâtit. La nouvelle rédaction de l'article 312-15 du Code de l'éducation nationale répare un oubli. Aujourd'hui, il omet de mentionner le fonctionnement de la vie démocratique et des institutions. Or, il s'agit bien d'un des objectifs premiers de cette discipline. La question de la formation des enseignants n'est pas abordée par ce texte, mais il semble primordial de mieux outiller les enseignants. La Commission de la Culture l'a rappelé à de nombreuses reprises qu'il s'agisse de la formation initiale ou continue. Je suis ainsi frappé que les épreuves du Capest d'histoire-géographie ne comportent aucune épreuve de EMC. Cette discipline impose, incombe pourtant, quasiment tout le temps à ses professeurs au collège. Du fait de son absence au CAPES, les INSPES ne sont pas incités à approfondir cet enseignement lors de la formation initiale. Il paraît essentiel que l'État joue pleinement son rôle de futur employeur et ainsi reprenne la main sur le contenu de la formation initiale des enseignants. Par ailleurs, la défense des valeurs de la République ne doit pas être laissée sous la seule responsabilité des professeurs d'histoire-géographie. Elle doit fédérer l'ensemble de l'équipe pédagogique, Nous devons être attentifs à la faire de leur transmission un projet partagé par l'ensemble de la communauté éducative. L'article 2 concerne la journée Défense et citoyenneté qui a connu les mêmes dérives. Elle était destinée initialement à être en rendez-vous obligatoire pour l'ensemble d'une classe d'âge avec les personnes participant à la défense du pays. Aujourd'hui, le temps consacré aux questions de défense et d'engagement est inférieur à trois heures. L'armée est consciente de la nécessité de faire évoluer cette journée et y travaille. Je rappelle que notre assemblée a adopté en juillet dernier, lors des débats sur la loi de programmation militaire, un amendement de notre collègue Henri Cabanel reprenant la rédaction de l'article 2 de ce texte. Il a d'ailleurs été maintenu dans la suite de la navette parlementaire, mais a finalement été censuré, car considéré comme un cavalier législatif. Cette proposition de loi vise également dans l'article 3 à faciliter l'insertion des jeunes suivis par les épides. Comme un certain nombre d'entre vous, j'ai eu l'occasion de me rendre dans un épide et y constater leur travail important pour accompagner des jeunes en grande difficulté vers l'insertion. Nous examinerons tout à l'heure un amendement de la Commission visant à préciser que l'accueil complémentaire de trois mois se fait dans la limite des places disponibles. En effet, selon les informations qui nous ont été transmises par le ministère du Travail, le taux d'occupation dans les épides serait de 90 à 95% selon les établissements. Je me réjouis de ce succès. En effet, la mission d'information avait souligné la nécessité de mieux faire connaître ces établissements. Ils souffraient d'une visibilité insuffisante parmi les dispositifs proposés aux jeunes sans qualification ni diplôme. Il me semble également important de renforcer le maillage territorial en lien avec les collectivités locales souvent demandeuses de l'installation d'un centre EPID. La directrice générale des EPID soulignait qu'une dizaine de départements avaient envoyé moins de Saint-Jeune en cinq ans en raison d'un maillage territorial trop faible. J'en viens maintenant aux articles 4 et 5 qui visent à moderniser le processus électoral. La société évolue. Aussi, je me félicite que le Sénat puisse débattre en séance d'une évolution de notre système électoral. Force est de constater que nous nous déplaçons de plus en plus. Et pour moi, il faut s'adapter. C'est ce que permet la double procuration. En ce qui concerne l'envoi dématérialisé de la propagande électorale, Je tiens à rassurer, il ne s'agit nullement de passer à une dématérialisation généralisée et obligatoire pour les électeurs. Un tel système aurait au contraire un effet pervers. 14 millions de Français ne maîtrisent pas le numérique. un certain nombre de nos concitoyens, notamment les plus jeunes, se disent intéressés par recevoir ces documents de manière dématérialisée. Nous sommes également tous conscients des difficultés logistiques pour distribuer dans un temps très court près de 48 millions de plis. Dans l'esprit des travaux de la mission d'information, la Commission a élargi la possibilité d'un envoi dématérialisé des documents de propagande électorale à l'ensemble des scrutins locaux ainsi que pour les élections européennes. Enfin, Ce texte vise à mieux reconnaître l'engagement des jeunes dans les mandats électoraux. Il est parfois difficile de concilier l'exercice du mandat avec le déroulement des études. Or, à la différence des élus salariés, il n'existe pas de garantie spécifique dans le code électoral pour les étudiants. Le Code de l'éducation ne prévoit pas non plus ce cas pour les aménagements d'études, alors même que d'autres engagements sont pris en compte, comme des engagements associatifs, militaires, civils ou encore lorsque l'étudiant travaille. Donc la Commission a réécrit l'article 6. Il lui a semblé plus judicieux de s'appuyer sur un dispositif déjà existant qui a fait ses preuves et qui répond aux besoins spécifiques des étudiants concernés. Par ailleurs, elle a étendu ce dispositif aux mandats nationaux et européens. Le rajeunissement de la classe politique concerne également nos assemblées. D'ailleurs, deux de nos collègues députés étaient étudiants au moment de leur élection. Donc mes chers collègues, cette proposition de loi s'inscrit dans un processus visant à guérir les fractures qui ont vu le jour entre les citoyens et les institutions. Enfin, permettez-moi en votre nom de saluer l'engagement de l'ensemble des élus locaux et notamment des maires qui sont présents à la tribune et qui sont un maillon essentiel de notre démocratie. Je vous remercie. Merci, merci chers collègues. Maintenant la parole dans la suite de la discussion générale est à madame Prisca Tevenot secrétaire d'état chargée de la jeunesse et du service national

Merci Monsieur le Président, Monsieur le Président de Commission, Monsieur le Rapporteur, Mesdames et Messieurs les Sénateurs. Je suis honorée de m'exprimer face à vous aujourd'hui pour la première fois à cette tribune depuis ma prise de fonction en tant que secrétaire d'État à la jeunesse, aux SNU et à la vie associative. ce secrétariat d'État que j'aime à qualifier de ministère du lien. Ministère du lien entre les jeunes eux-mêmes, entre les jeunes et la société au sein de la société elle-même. Ce lien est dans l'ADN de mon secrétariat d'État donc et des politiques publiques que je tiens à porter. Et je suis sûre qu'il sera au cœur de nos échanges ce matin sur un sujet aussi important que la citoyenneté socle de notre nation. Je souhaiterai ainsi remercier le groupe RDSE pour avoir mis à l'ordre du jour cette proposition complète, riche et constructive. Ce texte est effectivement le fruit d'un travail sénatorial transpartisan, extrêmement rigoureux, et le gouvernement en partage les constats. le goût des jeunes pour l'engagement, l'urgence de reconstruire la confiance entre citoyens et élus, le danger pour notre démocratie que représente la propagation des fake news sur les réseaux sociaux, et également le succès des dispositifs tels que le service civique. Ce texte, nous en partageons également pleinement la philosophie. Oui, l'engagement des jeunes est un véritable enjeu de cohésion nationale et nous devons aujourd'hui plus que jamais travailler à le renforcer. L'engagement, c'est le rappel que nous ne sommes pas simplement une somme d'individus mais bien une équipe, une équipe de citoyens engagés sous le même drapeau, partageant les mêmes valeurs, ces valeurs qui sont d'ailleurs en rappel sur les frontons de nos mairies et de nos écoles. Liberté, égalité, fraternité. Ces valeurs, nous devons plus que jamais les construire. Les construire dans le cadre d'une société résiliente, plus tolérante et plus unie. Et depuis six ans, nous devons l'appuyer également à l'endroit de notre jeunesse qui est au cœur de nos priorités. Notre jeunesse est aujourd'hui confrontée à la grande bascule, pour reprendre les mots du président de la République lui-même. Elle est confrontée à des défis importants, crise écologique, difficultés économiques et sociales, retour de la guerre en Europe, conflits sociaux et religieux, transformation numérique. Bref, face à cela, la jeunesse est unanime dans sa diversité. Elle ne veut pas être administrée, mais bien responsabilisée. Et en ce sens, oui, nous devons l'écouter et lui permettre de s'engager pleinement pour être actrice de son destin. Cette demande de responsabilisation, elle passe par l'émancipation citoyenne de chacun. Et nous devons l'entendre et la rendre audible. En 2019, nous avons lancé, avec Gabriel Attal, le service national universel. Dès lors, 90 000 jeunes ont pu y participer. Sur l'année 2024, nous allons ouvrir 80 000 places. Le SNU fait un pas de plus cette année avec le dispositif classe et lycée engagé. Il s'inscrira dans le cadre du parcours scolaire, dans le cadre d'un projet pédagogique annuel et sera déployé tout au long de l'année, aussi bien en classe de seconde qu'en première CAP. Nous avons à déjà dépasser nos objectifs de classe labellisée, preuve de l'engagement de l'entièreté du personnel éducatif. La moitié des classes qui ont répondu présentes pour cet appel à projet est issue des quartiers prioritaires de la ville. Cela permettra d'accroître la mixité sociale des jeunes volontaires au sein du séjour de cohésion SNU. Si le SNU, c'est effectivement, comme je viens de le rappeler, un séjour de cohésion de 12 jours, c'est aussi un temps d'engagement plus long à la Nation. J'ai annoncé vendredi dernier le lancement des brigades citoyennes SNU pour permettre aux jeunes volontaires de venir en aide aux collectivités locales et aux associations dans les territoires sinistrés par les intempéries partout en France hors temps scolaire et sur la base du volontariat bien sûr. Dès le lendemain, les premiers volontaires étaient déjà sur le terrain dans le Pas-de-Calais. Le service civique s'inscrit effectivement pleinement dans ce temps d'engagement plus long, qui est la phase 2 du service national universel. En 2024, nous ambitionnons 150 000 volontaires. Il s'agit du premier poste de dépenses de mon ministère, avec un budget annuel de 518,8 millions d'euros. Favoriser les échanges intergénérationnels et le vivre ensemble, c'est aussi l'objectif du service civique Solidarité Senior, lancé en 2021. Nos jeunes volontaires agissent pour lutter contre l'isolement de nos aînés tout en prévenant la perte d'autonomie et en participant à tisser une société plus solidaire. J'ai annoncé vendredi dernier le doublement du nombre de jeunes en services civiques Solidarité pour qu'ils puissent agir aussi bien en EHPAD qu'en résidence autonomie, avec un objectif d'intervenir auprès de 200 000 personnes âgées d'ici 2027. Pour reprendre les mots de votre rapport, redynamiser la culture citoyenne, c'est aussi permettre à nos jeunes de s'engager dans l'école de la citoyenneté que sont nos associations. Dès 2024, nous allons augmenter le FDA, le budget de fonds de développement à la vie associative qui permet de soutenir le fonctionnement des associations et plus particulièrement les petites structures. De 50 millions en 2023, nous allons ainsi passer à 70 millions en 2024. Comme je l'ai dit plus tôt dans nos sociétés, nous connaissons de profondes mutations et bien évidemment le secteur associatif n'y est pas hermétique. Il est donc de notre devoir, en plus de cet accompagnement financier, de les accompagner sur des démarches structurelles d'accompagnement autour de quatre grands axes simplification, reconnaissance, facilitation et bien évidemment accompagnement des acteurs eux-mêmes associatifs. J'en reviens maintenant au texte que nous examinons ce matin. L'article 1er propose de recentrer le contenu de l'enseignement moral et civique sur deux priorités, à savoir la connaissance des institutions françaises et européennes ainsi que la compréhension des grands enjeux internationaux, sociétaux et environnementaux. L'éducation morale et civique est un outil remarquable pour saisir le sens qu'ont les valeurs de notre République. À l'heure où les enjeux d'éducation aux médias sont de taille, la transmission d'une attitude réfléchie et éclairée vis-à-vis de l'information est un véritable besoin démocratique. C'est pour cela que le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, Gabriel Attal, a annoncé dès la rentrée 2024 que l'enseignement moral et civique serait renforcé à l'école et les heures seront doublées de la troisième à la cinquième. Nous partageons également la volonté de repenser le contenu de l'OMC. C'est la raison pour laquelle, à la demande du ministre, le conseil supérieur des programmes y travaillent en ce moment même et l'éducation aux médias et à l'information y sont bien évidemment pleinement intégrées. Les premières conclusions de ce travail seront attendues d'ici la fin du mois de décembre. Il me semble donc important de pouvoir attendre ces conclusions afin de modifier à nouveau la voie législative de l'EMC qui a déjà fait l'objet de nombreuses modifications ces dernières années. Par ailleurs, l'objectif de l'enseignement moral et civique ne peut se limiter à l'apprentissage de notre histoire, de nos valeurs, de notre culture politique, qui certes sont importantes, mais doit bien au-delà renforcer le principe de la République elle-même et ses valeurs dans une relation de confiance, comme cela a été rappelé juste avant. En somme, l'enseignement moral et civique doit être autant moral que civique. Par ailleurs, la fabrique du citoyen ne se limite pas à l'école. La Journée Défense et Citoyenneté constitue également une étape importante dans le parcours de citoyenneté. Elle doit retrouver sa vocation initiale de rendez-vous unique dans la vie d'un jeune avec les armées et avec tous ceux qui assurent la défense de notre pays. Cette journée doit être pensée comme une véritable expérience démocratique pour l'entièreté de notre jeunesse, qu'elle sensibilise aux notions d'engagement, de responsabilité et de fraternité. Dans cette perspective, le ministère des Armées travaille actuellement à la refonte de la journée de défense et de citoyenneté pour la recentrer sur ses missions premières, qui sont enseignés des enjeux et principes de la défense nationale, renforcer le lien entre les armées et la nation, et bien évidemment, accroître l'attractivité des métiers de défense et la volonté d'engagement de nos jeunes Français. Là encore, les travaux sont en cours, raison pour laquelle le ministère des Armées est réservé quant à l'article 2, non pas sur le fond, mais sur sa temporalité. La proposition de loi vise également à favoriser l'insertion des volontaires accueillis au sein des établissements pour l'insertion dans les emplois, les épides. Ce dispositif de seconde chance présente d'excellents résultats d'insertion au regard de la précarité des volontaires à leur entrée dans le dispositif. Le gouvernement est donc favorable à cet article sous réserve que l'amendement de réécriture du rapporteur soit adopté. Le gouvernement aimait être un avis défavorable sur les deux articles suivants qui concernent le processus électoral. En effet, le vote par procuration constitue une dérogation par principe du secret du vote. En 2021, dans le contexte de la crise sanitaire, le gouvernement avait fait le choix de déroger à ce plafond de dérogation. Le retour d'expérience nous montre qu'en réalité très peu d'électeurs se sont emparés de cette possibilité. Seuls 7% des mandataires étaient concernés par une double procuration et par ailleurs le gouvernement a assoupli le vote par procuration pour le rendre plus accessible. En effet, depuis le 1er janvier 2022, un électeur peut désormais donner procuration à un électeur inscrit sur une liste électorale d'une autre commune que la sienne. Concernant l'envoi dématérialisé du matériel de propagande électoral, si nous comprenons les enjeux de simplification et numérisation, l'inscrire dans le marbre de la loi semble prématuré, d'autant que cela nécessiterait une collecte de données de grande ampleur. En effet, aujourd'hui, seuls 25% des électeurs inscrits sur liste électorale ont renseigné leur adresse électronique à ce jour. Enfin, nos jeunes qui font le choix courageux de s'engager en politique, nous devons le tout faire pour leur faciliter la vie. Ils doivent pouvoir effectivement concilier leurs études avec leur mandat, qu'ils soient local, national ou européen. Je partage donc pleinement l'objectif de l'article 6 qui leur permet d'aménager leurs études tout en tenant compte de leurs obligations liées à leur mandat. Ce pantant est comme partagé, l'inscription dans le code général des collectivités territoriales ne semble pas parfaitement opportun. Mesdames et messieurs les sénateurs, au-delà de cette matinée, je souhaite que nous puissions poursuivre ce travail sur le renforcement du parcours citoyen tout au long de la vie. Nous devons continuer à avancer ensemble sur ce sujet d'une importance capitale pour notre pays, dans un esprit constructif. Faisons-le ensemble pour nos jeunes, et effectivement avec nos jeunes. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Gérard Laelek pour le groupe communiste républicain citoyen écologiste Kanaki. Et ce pour 4 minutes. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, tout d'abord, je souhaite saluer ici la volonté de cette proposition de loi qui répond à un objectif et à une nécessité que nous partageons, celle du renforcement de la culture de la citoyenneté. La création d'un statut pour les étudiants élus, ou encore le souci de vouloir ancrer dans notre temps le processus électoral en le modernisant, sont de bonnes avancées. L'enseignement moral et civique doit en effet s'attacher à transmettre les valeurs et les principes de la République qui fondent le pacte républicain. C'est une œuvre d'intégration républicaine et un devoir d'une institution scolaire vis-à-vis de chaque élève. Et disons-le, nous en avons grandement besoin. Je dis cela en pensant notamment à nos enseignants en général et à nos professeurs d'histoire et de géographie en particulier, aujourd'hui en grande souffrance, jusque dans leur classe. Oui, il faut instruire notre jeunesse du sens profond de notre République, car c'est à cette condition et seulement à cette condition qu'elle s'engagera elle-même pour la valoriser et pour la défendre. Mais, comme le disait si bien le grand Jaurès dans son discours de 1903 à la jeunesse, je le cite, « L'histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements, mais elle justifie l'invincible espoir. » Nous ne parviendrons donc pas à relever cet immense défi par quelques mesures symboliques, rappelant d'ailleurs par quelques aspects un retour aux heures glorieuses d'un passé où la journée scolaire commençait par la leçon de morale, écrite au tableau noir, et se clôturait parfois par une instruction civique à apprendre par cœur. Instituer la République, c'est proclamer que des millions d'hommes seront tracés eux-mêmes la règle commune de leur action, qu'ils seront conciliés la liberté et la loi, le mouvement et l'ordre. Or, cette PPL nous paraît moins ambitieuse précisément sur cette question de la liberté pleinement assumée. Sachons aussi de nous rappeler que notre République n'est pas né de la transposition de ce que fut la République romaine. Notre République est celle d'un grand peuple où il n'y a que des citoyens et où tous les citoyens sont réputés être égaux. Notre République, issue de la révolution, était aussi celle de la démocratie et du suffrage universel. C'était d'ailleurs une nouveauté magnifique et émouvante. C'est de cette nouveauté magnifique et émouvante qu'il faut instruire notre jeunesse. Non, nous ne préconisons pas de proposer à notre jeunesse un rêve décevant ni un rêve affaiblissant. Nous préconisons simplement d'enseigner à notre jeunesse le rêve éveillé d'une République en lui montrant contre toute menace et toute illumination qu'il faudrait en tout cas la défendre. En votant donc cette PPL, nous continuerons donc à nourrir cette grande ambition à enseigner et à faire partager à notre jeunesse. Je vous remercie de votre attention. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à madame Indique Girardin pour le groupe du RDSE Rassemblement Démocratique et Social Européen. C'est

très bien, j'oublie ma première feuille, ça se fait ça ? Monsieur le Président, excusez-moi. Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission de la Culture, Monsieur le rapporteur, Mes chers collègues, le groupe FDRDSE vous présente aujourd'hui une proposition de loi visant à renforcer la culture citoyenne, à savoir le lien entre le citoyen et les et les institutions. Elle comporte six mesures législatives d'ajustement qui se veulent être pratiques et pragmatiques. Henri Cabanel, son auteur, vient de vous la présenter. plusieurs années, voire des décennies, que nous inventons des dispositifs pour tenter de réaffirmer sans cesse, c'est que la citoyenneté et l'appartenance La France, pays des Lumières, mère patrie de la Révolution, pays des droits de l'homme et du citoyen, a permis de porter au regard du monde des valeurs telles que la laïcité, l'égalité, la fraternité ou encore la liberté. Elle fait face aujourd'hui à un problème majeur. Les héritiers de cette histoire, de ces combats, de ces victoires sont des tâches en méconnaissant totalement la valeur de cet héritage. Le constat de la perte de connaissance, cette compréhension de la construction de notre République, du fonctionnement de nos institutions et de la défiance envers la politique n'est pas nouveau. Mais même la volonté de vivre ensemble, de faire nation, est totalement en perte de vitesse. Alors cette citoyenneté, elle ne peut se construire qu'au quotidien, vous l'avez dit. Et nous pouvons même dire que cela doit être une construction perpétuelle à travers un parcours de vie. Mais encore faut-il en avoir les bases. Il faut dire que nous ne facilitons pas la tâche. À une époque où la synthèse est privilégiée face à nous avons, depuis des années, réussi à complexifier le contenu de nos apprentissages et la capacité d'accéder aux expériences citoyennes. C'est le cas des contenus de l'enseignement moral et civique qui aborde trop nombreux sujets en oubliant la priorité initiale, l'enseignement à la citoyenneté. C'est aussi le cas de la Journée Défense et Citoyenneté, pour rappel l'ex Journée d'Appel qui visait à remplacer le service militaire dans un contexte géopolitique complexe que nous connaissons aujourd'hui. Il n'est pas normal que la part de l'enseignement de la défense et de la sécurité se retrouve diluée dans un saupoudrage conduisant à des messages superficiels et peu audibles. La citoyenneté, c'est aussi l'expérience et l'engagement. Pour cela, les dispositifs sont nombreux. le conseil de la vie lycéenne, les éco-délégés, le service national universel, le service civique, les VIA, les VIE, les conseils municipaux des jeunes, les multiples conseils d'administration étudiants. Alors pourquoi ne sont-ils pas suffisamment plébiscités ? La réponse est sans doute liée au manque d'accompagnement et aux facilités données à tous les jeunes d'y accéder. La réponse est également dans les dispositifs qui sont insuffisamment complémentaires les uns des autres, entre apprentissage initial et pratique, et encore un sujet, la valorisation de cet engagement. J'ai entendu, Madame la Ministre, ce que vous souhaitez mettre en place, ce que souhaite mettre en place le ministre de l'Education nationale ou encore de la Défense. Et j'espère qu'on pourra répondre effectivement à toutes ces questions. Mais il faut aller vite, très vite. Alors être citoyen, c'est aussi faire des choix politiques. Ces choix passent par le vote et par la participation à la décision, la progression de l'abstention. On sera nombreux à le dire durant toutes les échéances ou pour toutes les échéances électorales. C'est un élément qui nous oblige aujourd'hui à réagir, à réagir rapidement, permettre par exemple la double procuration durant le processus électoral, recourir à l'envoi électronique des professions de foi. Ce sont des mesures de bon sens que le groupe RDSE vous propose aujourd'hui, avançant. Voter cette loi c'est aussi favoriser la participation des jeunes à la vie démocratique en accordant la protection aux étudiants, exerçant un mandat d'élu local ou encore accompagner les jeunes sans diplôme dans la consolidation de leur insertion en prolongeant l'accompagnement des épides. Et un exemple sans doute à suivre ce qu'on appelle dans les territoires outre-mer le service militaire adapté où on est allé très loin sur l'engagement. L'outre-mer peut inspirer la nation davantage. Alors, c'est avec beaucoup de fierté que notre groupe propose et soutient cette proposition de loi qui, je l'espère, sera aussi votée favorablement par l'ensemble des sénateurs des sénateurs ici présents sur l'ensemble des bancs. Bien entendu, je ne peux pas conclure sans saluer mes deux collègues Henri Cabanel à l'initiative de cette loi, Bernard J'ai l'air qu'il y en a été 100 rapporteurs et enfin je veux dire que je pense intimement que ce travail devra se poursuivre par une matérialisation d'un parcours citoyen se déroulant tout au long de la vie et ce qui nous permettra de consolider un socle civique commun. Voilà, ce parcours prendra la forme, je l'espère, d'un jour d'un passeport qui viendra sceller les droits et les devoirs des citoyens français

Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission de la Culture, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues, La culture citoyenne est cruciale pour le renforcement du lien entre les citoyens et les institutions, une préoccupation que nous partageons pleinement au sein du Groupe RDPI. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui découle des recommandations émanant de la mission d'information « Comment redynamiser la culture citoyenne ». Cette mission avait pour objectif d'explorer les fondements actuels de la culture citoyenne et de trouver des moyens de renforcer l'adhésion des citoyens à un projet commun reposant sur des références partagées. La mission d'information a identifié cinq étapes essentielles pour permettre aux citoyens de s'inscrire dans un projet collectif à travers un parcours citoyen tout au long de la vie. Ces étapes comprennent l'école, la journée, défense et citoyenneté, les dispositifs d'insertion sociale, l'engagement citoyen et les élections. La PPL concentre ses efforts sur la formation de la citoyenneté, qu'elle entend améliorer, les modalités électorales qu'elle entend moderniser et l'engagement des jeunes dans les mondes à locaux qu'elle entend faciliter. Permettez-moi de souligner les principales dispositions de cette proposition de loi que je considère comme des avancées significatives. Tout d'abord, la révision de l'enseignement moral et civique porté par l'article 1 vise à recentrer son contenu, notamment sur une meilleure connaissance du fonctionnement des institutions françaises et européennes. Cela représente un pas essentiel vers la formation des citoyens informés et engagés. L'article 2, relatif à la journée Défense et citoyenneté, propose un recentrage sur des thèmes spécifiques tels que la défense, la sécurité, les métiers accessibles aux jeunes qui voudraient servir leur pays. L'orientation des jeunes en difficulté et la présentation des différentes formes d'engagement. Cela contribuera sans aucun doute à une meilleure compréhension des enjeux cruciaux auxquels notre nation est confrontée. L'article 3 propose une prolongation de trois mois du contrat d'accompagnement au sein de l'établissement pour l'insertion à l'emploi, offrant ainsi aux jeunes volontaires une période supplémentaire pour s'adapter, se développer et faciliter leur intégration dans la société. Si le rétablissement à l'article 4 de la double procuration peut représenter pour certains une avancée vers une plus grande participation citoyenne au scrutin, une partie des membres de notre groupe est défavorable à la double procuration compte tenu de l'importance du caractère dérogatoire du vote par procuration et du principe du secret du vote. Par ailleurs, la transition vers la propagande électorale électronique reflète une volonté d'adapter nos pratiques démocratiques aux évolutions technologiques. Matérialisée dans un cinquième article, elle entend offrir aux électeurs la possibilité de choisir le format qui leur convient le mieux, voulant favoriser ainsi une participation accrue. Est-ce si certain ? Permettez-moi de rappeler le risque de marginalisation de ceux qui n'ont pas accès à Internet ou qui ne sont pas familiers avec les nouvelles technologies. D'après l'INSEE, ça a été répété tout à l'heure, 15,4% des personnes de 15 ans ou plus résident en France étaient en situation d'électronisme. Enfin, la création du statut de l'élu étudiant à l'article 6 est une mesure qui mérite d'être saluée. Elle reconnaît l'engagement des jeunes étudiants dans la vie politique locale, régionale et départementale en leur garantissant des aménagements nécessaires. Cependant, je tiens à exprimer un regret partagé par bon nombre de sénateurs de notre groupe. Alors que la lettre de saisine du Conseil supérieur des programmes l'invitait à dépasser le cadre de l'enseignement du fonctionnement des institutions, n'aurait-il pas été nécessaire d'attendre la diffusion de ces travaux pour éclairer encore plus cette PPL ? Dans cette lettre, je le rappelle, le ministre commande la rénovation des programmes de l'enseignement moral et civique depuis le cours préparatoire jusqu'à la classe terminale. Il exprime une ambition renouvelée pour l'enseignement moral et civique et souligne son rôle crucial dans l'information des élèves en tant que citoyen éclairé. Cette lettre souligne également l'importance de transmettre une conception de la citoyenneté, mettant à la fois l'accent sur l'autonomie du citoyen et son appartenance à une communauté politique. Ceci inclut la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que la lutte contre toutes les formes de discrimination. De plus, la connaissance des institutions de la République et de l'Union européenne est mise en avant. Dans cette logique, elle annonce déjà le doublement de l'horaire de l'enseignement moral et civil en cycle 4. Elle l'enrichit avec des modules d'éducation en médias à l'information, notamment dans l'espace numérique et sur les réseaux sociaux, avec un seul objectif, l'apprentissage au discernement. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, bien que cette proposition soit porteuse d'une vision ambitieuse pour la culture citoyenne, sa non articulation avec la lettre de mission n'est pas sans nous interroger. Par ailleurs, comme nous l'évoquions précédemment, les articles 4 et 5 soulèvent de nombreuses interrogations ne permettant pas à notre groupe d'avoir un vote unanime. Je vous remercie. votre discours. La parole est maintenant à monsieur Adelzian pour six minutes pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Merci madame. Merci madame. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le Rapporteur, chers collègues, nous est donné l'opportunité aujourd'hui de débattre d'un concept ô combien essentiel pour le ciment de notre République, la citoyenneté. La citoyenneté en France qui s'est forgée dans les luttes et les aspirations de notre peuple au cours des siècles, inspirée de l'Antiquité, mûrie Par les lumières concrétisées avec la révolution de 1789, souvenons-nous quand même que ce concept de citoyenneté revêtait autrefois un caractère d'exclusion pour l'ensemble des femmes et pour les hommes qui ne pouvaient s'acquitter du sens. Je pense à la classe laborieuse qui, à la suite d'une longue lutte politique, a dû attendre 1848 avant que le vote bascule du scrutin sensitaire à celui dit universel, et encore, imparfaitement universel, car celui-ci ne le deviendra pleinement que près de 100 ans plus tard à la suite d'une lutte encore plus longue et âpre avec le vote des femmes en 1945. La construction européenne apportera sa pierre à l'édifice, à la citoyenneté en 1992 avec la citoyenneté européenne et le traité de Maastricht. Aujourd'hui, en 2023, ce combat, cette lutte continue et la citoyenneté est bien plus qu'un simple statut administratif. Elle est confrontée à de nouveaux défis, à de nouveaux enjeux que ce débat aujourd'hui nous permet de discuter. Au concept d'individu citoyen, au sens d'un individu qui détient des droits, des devoirs et participe à la vie politique de la cité, à la recherche d'un idéal commun tend à se substituer lentement celui de l'individu consommateur, délaissant la production d'idées, de convictions, d'engagement, de solidarité au profit d'un intérêt tourné quasi exclusivement à celui de sa propre consommation de biens et de services. La mondialisation, les crises environnementales, les avancées technologiques remettent en question ce rôle en tant que citoyens. L'abstention interroge quand on faille de notre modèle actuel de citoyenneté, révélateur d'une partie des abstentionnistes d'un désintérêt complet pour la politique dans ses composantes, une autre partie ne considérant plus que le vote assure un débouché démocratique et donc s'organise en conséquence avec d'autres modes d'action à l'image du mouvement des Gilets jaunes. Dans le passé, notre modèle de citoyenneté a su évoluer, comme je le disais, s'adapter aux époques dans lesquelles ces acteurs évoluent. L'enjeu est majeur, et nous en parlerons aujourd'hui, c'est l'adhésion aux valeurs de la République, d'égalité, de liberté, de fraternité, qui ne peuvent être mises en péril. C'est le sens de cette proposition de loi, qui de toute évidence, si elle n'apporte pas de changement substantiel ou d'avancée significative dans la promotion de la citoyenneté, nous la saluons, et nous saluons les propositions portées toutes issues des recommandations d'un rapport d'information. le mérite de l'initiative et la volonté de contribuer à ce débat de notre collègue Henri Cabanel. Et si la question se pose de savoir si cette proposition noire répond aux défis contemporains de la citoyenneté, malheureusement elle sera imparfaite, ne sera pas forcément positive, car ces enjeux actuels, comme je le disais, nécessitent une approche plus ambitieuse et des mesures plus substantielles pour renforcer l'engagement citoyen. Malgré cela, le groupe socialiste reconnaît les avancées proposées par cette loi. Ces mesures vont avec le présent article n°1 dans le sens d'un enseignement moral et civique opérationnel qui replace les enjeux institutionnels au cœur de celui-ci. permettre aux plus jeunes apprentis citoyens d'apprendre au mieux les outils démocratiques qu'ils auront en leur possession à la majorité. L'article 4, qui pérenniserait la double procuration mise en place lors de la pandémie de Covid-19, facilite les conditions de participation matérielle des électeurs ou scrutins, mais nous appellerons également une vigilance forte dans sa mise en oeuvre opérationnelle pour éviter tout usage. Enfin, l'article 6, le plus ambitieux, favorise la participation des jeunes à la vie démocratique et c'est le cœur du sujet. Ils prévoient des aménagements dans le déroulement de leurs études, dans le cadre d'étudiants dépositaires d'un mandat municipal, départemental ou régional. Car cet être citoyen, c'est aussi être en capacité d'avoir des droits et en capacité de les utiliser. Et nous nous réjouissons qu'au stade de la Commission, il est étendu aux mandats nationaux et européens. En tant que partisans du progrès et de l'égalité, nous ne pouvons ignorer les opportunités de ce texte, tendant à renforcer la pratique citoyenne, même si, je le répète, elle reste modeste pour un certain nombre de points. Pour aborder de manière plus approfondie les enjeux de la citoyenneté, il serait dès lors impératif dans les années à venir, ici même, d'explorer des pistes complémentaires. Nous devons envisager des réformes éducatives plus audacieuses, intégrant davantage les questions de citoyenneté, de participation civique dans les programmes scolaires. De plus, une réflexion sur la représentativité des institutions et la participation citoyenne directe pourrait être envisagée pour renforcer la légitimité démocratique. Hier, lors de notre niche, la proposition de loi constitutionnelle de notre collègue Yann Chantrelle visant à faciliter le déclenchement du référendum d'initiative partagée a été examinée, malheureusement rejetée, mais elle allait dans ce sens et je regrette que nous n'ayons pu l'adopter. Enfin, dans un monde de communication et d'information omniprésent, où il devient de plus en difficile de traiter et d'analyser, nous devons également, et j'insiste sur ce point, nous attaquer à la désinformation et promouvoir une éducation aux médias et à la pensée critique. Ainsi, le groupe socialiste fidèle à ses principes et à son engagement envers le bien commun votera en faveur de la présente proposition de loi. Nous considérons que même les petits avancées, les petits pas peuvent être les premiers pas vers des changements plus importants, plus majeurs. Cependant, nous appelons nos collègues à ne pas perdre de vue l'urgence d'une réflexion plus approfondie sur les défis actuels de la citoyenneté dont nous avons pu débattre hier encore. Je vous remercie de votre attention. Merci chers collègues. La parole est désormais à madame Sabine Drexler pour le groupe Les Républicains pour 8 minutes.

Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, depuis 1789, nous sommes tous reconnus comme des citoyens et nous faisons partie d'une même nation, une nation démocratique où la souveraineté appartient au peuple qui est appelée à donner son avis quant aux décisions qui le concernent en s'exprimant à travers son vote. Aujourd'hui, nous vivons une profonde crise démocratique qui se manifeste notamment par une lente érosion de la participation à toutes les élections. L'abstention est même devenue ce que d'aucuns appellent le premier parti de France, avec un record atteint en 2021 lors des élections départementales et régionales, avec seulement un tiers de votants. Cet état des lieux interpelle, inquiète, évidemment, et au Sénat, nous réfléchissons aux causes de ce phénomène, mais aussi aux solutions à apporter pour réenchanter la politique et renouer les fils de la confiance entre les citoyens et leurs représentants. Faut-il pourtant être défaitiste ? Je ne le pense pas et il ne le faut pas. Car les citoyens, en fait, ne demandent qu'à y croire. Cet état des lieux est la traduction d'un mécontentement, celui d'électeurs qui n'y croient plus, mais aussi le signe d'une méconnaissance des institutions du haut-réforme successif qui ont rendu illisible pour les citoyens le paysage institutionnel de notre pays. Car effectivement, et c'est regrettable, le problème majeur du système d'administration français est l'incohérente et complexe répartition des compétences entre les collectivités territoriales entre elles et avec les services de l'État eux-mêmes organisés sur plusieurs niveaux. Périodiquement, des lois cherchent à rationaliser la distribution des compétences avec comme seul résultat de compliquer encore davantage le paysage. C'est émiettement des responsabilités pour gérer des affaires qui sont fortement interdépendantes à d'innombrables défauts dont l'opacité du système pour les citoyens, ce qui contribue à leur démotivation lors des élections et à leur méfiance à l'égard d'un système incompréhensible avec ses multiples acteurs aux responsabilités mystérieuses. Il est également le fruit d'une longue dégradation du débat public, une dégradation qui a remplacé la parole par l'invective. Cet essoufflement démocratique, nous pouvons l'endiguer. par des mesures, excusez-moi, comme celles qui nous sont aujourd'hui proposées dans cette proposition de loi qui est une première étape, une étape qui devra en appeler d'autres, pour continuer à retisser les fils de la confiance perdue. Si je devais qualifier le texte dont nous allons débattre aujourd'hui, je proposerais trois mots. Recentrer, faciliter et encourager. Pourquoi recentrer ? L'école et l'éducation sont les terreaux qui forgent les citoyens de demain. Mais pour cela, faut-il encore que l'instruction civique dispensée dans les classes de notre République soit comme autrefois une discipline à part entière et non un enseignement strapontin, comme le qualifie très justement le rapporteur Bernard Fialer. Le MC est aujourd'hui un fourre-tout qui a perdu de vue ses objectifs initiaux et qu'il faut pouvoir recentrer sur ses fondamentaux l'esprit républicain, les valeurs démocratiques mais aussi la morale. Il est également essentiel, fondamental même, de former les élèves à la connaissance des institutions, des mécanismes de vote et des élections, au fonctionnement administratif, au fonctionnement de la justice et des instances de gouvernement. Cette refonte devra passer par des supports pédagogiques repensés, repensés, recentrés et simplifiés. La journée de jeunesse et citoyenneté quant à elle est certes une occasion de nouer un contact direct avec les militaires, de sensibiliser aux enjeux mondiaux et nationaux de défense dans un monde où les conflits armés se multiplient. Mais il y a une vraie nécessité aujourd'hui de recentrer le contenu de cette journée sur les enjeux de sécurité et de défense, ainsi que des différentes formes d'engagement ce qui contribuera à faire de nos jeunes des citoyens responsables et éclairés capables de réfléchir et de penser par eux-mêmes, d'avoir un avis personnel pour qu'ils ne se laissent pas manipuler car c'est l'ignorance ou le déni qui font le lit des guerres en mobilisant les plus influençables autour de causes qui ne sont pas les leurs. Et pourquoi faciliter ? Les établissements pour l'insertion dans l'emploi à les épides sont des structures qui, depuis 18 ans, font la preuve de leur performance. Avec près de 50 000 jeunes sortis des épides et un taux d'insertion dans l'emploi de plus de 40%, c'est une solution qu'il faut continuer à développer et à soutenir. En cela, la proposition qui est faite par le rapporteur d'ouvrir la possibilité de prolonger la durée d'hébergement et l'accompagnement des jeunes travailleurs de trois mois est sans nul doute une excellente chose dans le contexte actuel où l'accès au logement est l'une des principales difficultés rencontrées par les jeunes travailleurs. J'en arrive aux mesures qui concernent le processus électoral et l'amélioration de la formation délivrée aux électeurs. Là encore, et pour commencer par ce qu'il y a de plus simple, je pense qu'il nous faut que nous pouvons cadérer aux principes et à la nécessité de faciliter les démarches pour inciter les électeurs à voter. Faciliter, c'est aussi encourager. En ouvrant la possibilité de la double procuration, nous répondons aux attentes exprimées par les citoyens. De même, ouvrir la possibilité de diffuser la propagande électorale par voie électronique me semble être une réponse qui devrait permettre de faire repartir la participation électorale à la hausse. C'est une attente forte, notamment des jeunes générations et de celles qui sont le plus éloignées du vote dans sa forme traditionnelle, telle que nous l'avons nous toujours connue. Une technique de vote directe qui ne nécessitera pas de se déplacer et qui permettra en outre et à terme d'éviter le gâchis qui nous questionne tous, celui de milliers de tonnes de papiers et d'encre, sans même parler de l'organisation logistique qu'elle implique avec la mise sous pli chronophage par les préfectures ou les collectivités et des difficultés liées à sa distribution que nous avons notamment pu constater lors des derniers scrutins. En mettant en place un système mixte d'envoi de la propagande électorale par voie électronique et écrite, nous ne pourrons que davantage inciter les électeurs à voter. Et enfin, pourquoi encourager ? Nous savons que les jeunes générations se détournent de plus en plus de l'engagement associatif ou politique faute de temps, mais aussi parce qu'il est difficile pour eux de concilier un tel engagement avec leurs études ou le début de leur carrière dans la vie active. à l'heure où l'engagement politique est de plus en plus chronophage et complexe et où nous vivons une crise profonde des vocations qui se traduit en particulier par un record jamais connu de démission de maires et d'élus locaux, je me réjouis que l'on puisse ouvrir la voie à ce droit particulier très incitatif pour les étudiants et je ne doute pas qu'ainsi nous inciterons à nouveau une partie de nos jeunes à s'engager dans la vie locale. Et pour finir, chers collègues, Il me semble que sur ces sujets il nous faut dépasser les clivages politiques car la santé de notre démocratie est en jeu. Cette première étape, je l'espère, en appellera d'autres et en tout état de cause poursuivons ensemble cet objectif ambitieux de proposer des solutions et de souciter à nouveau l'envie, l'envie de s'exprimer en sachant être entendu, l'envie de s'engager en sachant que sa mobilisation a de la valeur et est reconnue en tant que telle et surtout l'envie et la fierté d'être en toute connaissance de cause un citoyen français. Je vous remercie. Merci beaucoup madame la sénatrice. La parole est maintenant à madame Laura Darkos pour le groupe Les Indépendants. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues, permettez-moi aussi de saluer dans les tribunes mon ami Pierrick Courillot, qui est un élu avec des handicaps lourds. Il va me suivre toute la journée, mais c'est un élu extrêmement dynamique et il montre qu'on peut bien évidemment apporter beaucoup de choses dans sa vie municipale en ayant tous ces handicaps. Pierrick, je te salue. En juin 2022, Henri Cabanel, que je salue ici, rapporteur de la mission d'affirmation sur la redénonisation de la culture citoyenne, à laquelle j'ai été heureuse de participer, ouvrait la voie de nouvelles mesures visant à restaurer le lien entre les citoyens et les institutions. Les différents articles que nous examinons aujourd'hui constituent la transcription de plusieurs préconisations législatives issues du rapport d'information. Pour cette raison, je félicite l'auteur de ce texte ainsi que son rapporteur pour leur excellent travail. Cette proposition de loi apporte des réponses concrètes au désengagement démocratique des Français dont témoignent à intervalles réguliers les taux d'abstention lors des élections locales et nationales. Nous savons à quel point nos concitoyens connaissent mal le fonctionnement de nos institutions et sans désintérêt. C'est d'autant plus vrai pour les jeunes qui, pourtant, reçoivent un enseignement moral et civique relativement dense tout au long de leur cursus scolaire. Nous sommes tous préoccupés par le délitement progressif de nos valeurs communes qui s'accompagne d'un fossé grandissant entre l'élu et le citoyen. Une certaine fatigue républicaine s'est emparée de notre pays. Ce texte permet de traiter le mal à la racine en formulant des propositions pertinentes et réalistes. Dans la droite ligne des conclusions de la mission d'information, deux articles de cette proposition loi visent à moderniser le processus électoral. Je cellule l'introduction de la double procuration et la création d'un cadre mixte de diffusion de la propagande électorale. Il permettra aux candidats de transmettre leur profession de foi numérisée aux électeurs qui en font la demande. Cela représente une vraie avancée sur le plan écologique, bien sûr, mais aussi sur le plan logistique, tant les services de diffusion postale sont engorgés en période électorale. Il arrive même que dans certaines communes, les habitants reçoivent la propagande électorale après les élections, ce qui est un non-sens démocratique. Il s'agit également de rapprocher les plus jeunes de la vie citoyenne. La mission d'information, invité à réduire et clarifier les notions abordées en classe d'enseignement moral et civique. Le texte propose de recentrer le contenu des enseignements sur l'étude des institutions françaises. Cette proposition est judicieuse compte tenu du manque de cohérence qui caractérise le programme actuel de l'EMC dont les objectifs sont pour le moins disparates. De la même manière, la création d'un statut d'élu étudiant est une excellente mesure. Nous devons encourager ces jeunes vocations dédiées au service de l'intérêt général. En cette semaine consacrée aux maires de France, je tiens à saluer tout particulièrement les plus jeunes d'entre eux. Si la proposition de loi ne propose pas de disposition spécifique sur le service national universel, je voudrais néanmoins l'évoquer, car il s'agit incontestablement d'un moyen de valoriser la citoyenneté, de renforcer la cohésion sociale et de faire découvrir le sens de l'engagement. Le séjour de cohésion permet en effet pendant 12 jours un brassage social qui n'existe plus depuis la fin de la conscription. Quant à la mission d'intérêt général, elle offre aux volontaires du SNU la possibilité de se mettre au service des autres, dans une logique désintéressée. Je salue à ce sujet l'initiative prise par madame la secrétaire d'État, chargée de la jeunesse et du service national universel, qui a annoncé le déploiement des brigades citoyennes SNU auprès des collectivités territoriales et des associations venant en aide aux habitants victimes des inondations dans les Hauts-de-France. Le SNU est donc le bon support pour faire grandir les jeunes et les aider à se réaliser en tant que citoyens. C'est pourquoi je suis favorable à son extension à l'ensemble d'une classe d'âge, même si je ne méconnais pas les défis budgétaires, logistiques et d'organisations immenses que cette extension impliquerait. Dans les médias, nous pourrions dégager quelques marges de manoeuvre financière avec un peu de bon sens en affectant les jeunes volontaires à proximité de leur domicile dans le périmètre régional. Néanmoins, comme le souligne très justement la mission d'information, la saisine du Parlement sera indispensable pour mettre fin à l'ambiguïté du SNU et trancher enfin sur sa nature militaire ou civique, volontaire ou obligatoire. En tout état de cause, la proposition de loi qui nous est soumise est pertinente et le groupe Les Indépendants lui apportera son soutien. Je vous remercie. Merci beaucoup Madame la Sénatrice. La parole est maintenant à Monsieur Jean Ingret pour l'Union centriste.

M. le Président, Mme la Ministre, M. le Président de la Commission, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à saluer, comme de nombreux interlocuteurs avant moi, à féliciter Henri Cabanel pour sa proposition de loi, ainsi que le travail de Stéphane Piednoir suite à l'élaboration de sa mission d'information sur le sujet de la culture citoyenne. Comme j'ai déjà pu l'exprimer en commission, les sénateurs du groupe union centristes sont intimement convaincus que cette proposition de loi va dans le bon sens. Personne ici ne peut contester qu'un fossé se creuse entre les élus et les citoyens. Le rapport de la mission d'information fait par notre collègue est particulièrement éloquent. Cette proposition de loi vient donc apporter une traduction législative aux recommandations de cette mission. Sur la réforme du code de l'éducation d'abord, nous saluons la volonté de réforme de ce code si complexe pour y faire apparaître une formation aux valeurs de la République dans le cadre de l'enseignement civiques civiques et morales. Nous ne pouvons en effet que déplorer la mauvaise connaissance de nos institutions par les plus jeunes, mais également par une part de plus en plus importante de la population, perdue entre les compétences des différents échelons territoriaux et le rôle des différentes institutions. Sacraliser un minimum de pédagogie sur nos institutions et sur le principe de laïcité est une réelle avancée. Nous pouvons faire le voeu que les plus jeunes seront informés du rôle de chaque élu et plus ils participeront au scrutin. Introduire une réforme de la Journée Défense et Citoyenneté est également une bonne chose. Nous partageons la vision d'Henri Cabanel sur le fait qu'un recentrage des thématiques abordées lors de cette journée est absolument nécessaire tant on voit l'éparpillement des sujets traités sur une seule journée. Les sensibilisations sur le thème de l'égalité femmes-hommes ou sur le don d'organes existent au sein des établissements scolaires. Recentrer la journée défense et citoyenneté pour véritablement promouvoir l'engagement au sein des forces armées. armées. Des réserves ou encore des sapeurs-pompiers est une bonne chose. Cela pourra naturellement susciter de nouvelles vocations. Cette proposition de loi va permettre aussi, en tout cas on l'espère, de réformer le processus électoral avec le retour à la double procuration. Nous savons que cela est faisable. Fort de la mise en place faite lors des élections départementales et régionales de 2021, la double procuration pourrait utilement contribuer à diminuer l'abstention, notamment chez les plus jeunes. Par exemple, s'ils sont en études loin du domicile familial ou s'ils sont encore inscrits sur des listes électorales éloignées de leur lieu d'études, le recours aux doubles procurations pourrait faciliter le vote par les familles ou par les amis. Toujours pour les plus jeunes, mais aussi pour l'ensemble du corps électoral, avoir recours à un envoi dématérialisé de la propagande électorale est une démarche encourageante. Nous ne sommes pas certains qu'arrêter les envois par courrier soit pertinent à ce stade. Et ce n'est d'ailleurs pas l'objet de cette présente proposition. Un envoi par mail de la propagande serait un bon complément à l'envoi postal. Les documents arriveraient des validations par la commission de propagande par courriel, gagnant ainsi du temps sur les opérations d'impression, de missoupli et d'acheminement postal. Les électeurs pourraient ainsi avoir davantage de temps pour prendre connaissance des différentes candidatures, des programmes, prendre aussi quelques heures d'avance sur le scrutin pour s'intéresser aux différents modes électoraux comme c'était le cas lors des élections de 2021. Cette mesure elle aussi est encouragée car elle permet une meilleure information des citoyens et éventuellement d'amorcer une réorganisation de la diffusion de la propagande électorale. Innovation aussi dans cette proposition de loi que la création d'un statut d'élu étudiant sur un modèle de l'étudiant salarié. Ce statut apporterait des facilités aux étudiants disposant d'un mandat électif pour mieux combiner études et mandats via des aménagements dans l'organisation du temps d'études et des examens. On imagine aisément que de jeunes qui cherchent à s'engager dans des mandats électifs, s'ils sont encore en études, trouveraient beaucoup plus de facilité pour être élus, en cause notamment l'éloignement géographique entre le lieu d'élection et le lieu d'étude sur lequel il est difficile d'agir, mais aussi sur l'investissement en temps. Ce nouveau statut pourrait ainsi apporter des solutions à cette seconde problématique et permettre à des étudiants de pouvoir être candidat aux élections et ensuite exercer leur mandat. Comme vous l'avez compris, mes chers collègues, l'ensemble des sénateurs de l'Union centriste soutient les différentes mesures proposées dans cette proposition de loi et nous encourageons vivement nos collègues à aller de l'avant sur ces différentes mesures. Je vous remercie. Merci chers collègues. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à madame Mathilde Olivier pour le groupe écologiste Solidarité et territoire. À vous madame. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je rejoins le constat que pose cette proposition de loi. Notre pays est plus fracturé que jamais. Les explications et causes diverses ne sont pas simples à appréhender. Elles nécessitent forcément nuance et réflexion. Les crises à répétition, les difficultés économiques ou sociales, l'exemple arrêté même de la classe politique, sont tant de raisons qui peuvent expliquer ce fossé entre les citoyens et la citoyenneté. Nous, chez les écologistes, nous sommes convaincus que le vivre ensemble doit se conjuguer au faire ensemble. Nous devons travailler la question du lien, du lien dans le travail, dans nos métiers, du lien dans nos vies, dans nos villes et dans nos villages. Je souhaite saluer l'esprit de cette proposition de loi qui veut apporter des réponses à notre principe fondamental du faire société. Un principe qui va mal, qui se trouve dans une impasse aujourd'hui. Cependant, je voulais vous alerter sur certains points. Vous évoquez à plusieurs reprises la forte fluctuation législative ces dernières années au sujet des premiers articles de la proposition. Je m'interroge alors sur la logique à notre tour de légiférer encore et encore sur le cours enseignement moral et civique et sur la journée défense et citoyenneté. Pour l'enseignement moral et civique, nous restons convaincus que c'est la liberté d'enseignement de nos professeurs qui permettra la meilleure compréhension et le meilleur apprentissage de la citoyenneté. faisant confiance au corps enseignant et apportant lui les moyens pour faire de ce cours une matière centrale dans le quotidien des élèves. Pour la journée défense et citoyenneté, je regrette que les mentions liées à la lutte contre les préjugés sexistes et contre les violences physiques, psychologiques ou sexuelles aient été supprimées, alors que tous les jeunes n'ont pas accès à de tels modules et que ces questions sont primordiales aujourd'hui. Nous accueillons positivement les articles sur l'envoi électronique de la propagande électorale, qui est un tournant que nous ne devons plus hésiter à prendre. Nous nous rappelons toutes et tous du fiasco de la distribution des documents électoraux lors des dernières législatives. Cette situation ne doit pas se reproduire. Pour les Françaises et les Français de l'étranger, nous fonctionnons d'ailleurs de cette manière depuis déjà des années. Cela permet de réduire considérablement les risques de dysfonctionnement, mais aussi l'empreinte carbone des impressions papier. Ces dispositions aient et doivent bien sûr rester facultatives et ne pas aggraver la fracture numérique. De même, au sujet de la double délégation de vote, cet usage fonctionne et a fait ses preuves preuves pour nous, Françaises et Français de l'étranger, et nous voyons positivement cette généralisation. Il reste nécessaire de bien communiquer sur cette possibilité et sur le processus d'établissement de procuration. Une des grandes préoccupations de notre démocratie concerne l'abstention affolante. Une société où tant de personnes ne votent pas, c'est une société malade. Aux dernières élections présidentielles, 42% des 18-24 ans ne se sont pas rendus aux urnes. Aux dernières élections législatives et municipales, plus de 70% des jeunes se sont abstenus de voter. Je me félicite que cette proposition de loi s'engage à mieux reconnaître l'engagement des jeunes dans les mandats politiques. C'est l'un des leviers pour lutter contre l'abstention. Concilier vie d'engagement, vie d'études et vie personnelle reste pour de nombreux jeunes citoyens un véritable obstacle. Le taux de maire de plus de 60 ans a atteint 55,3% en 2020. Le temps est un critère non négociable dans la démarche d'engagement. Sauter le pas de la représentativité est encore beaucoup trop compliqué pour les jeunes citoyens. Mais il y a de l'espoir dans les conseils municipaux, régionaux, à l'Assemblée, au Sénat, des jeunes passent le pas. Leur permettre de libérer du temps pour leur mandat, qu'il soit locaux ou nationaux, c'est une bonne chose. Mais demain, il faudra évidemment aller encore plus loin. Mes chers collègues, combattre le frein de l'engagement politique des jeunes, c'est aussi leur laisser la place et les accompagner dans cette démarche. C'est par l'action qu'on engrange expérience et confiance. Faire et vivre en société, c'est favoriser l'engagement de toutes et tous, quel que soit l'âge, le genre ou le milieu social. La jeunesse est notre pilier, donnons-lui sa chance. Sur l'ensemble du texte, la démarche nous semble aller dans le bon sens. C'est pour cette raison que le groupe écologiste Solidarité et territoire votera en faveur de cette proposition de loi tendant à renforcer la culture citoyenne. Merci, merci chers collègues. La discussion générale est désormais close. Nous passons à la discussion du texte de la Commission. Et je suis saisi d'une demande de parole à l'article 1er par le président Pierre Ousoulias. Merci Monsieur le Président, merci, bonjour Madame la Ministre. Chers collègues, je me félicite de cette nouvelle rédaction de l'article L312-15 du Code de l'éducation qui est sobre, efficace et qui, je pense, sera beaucoup plus facile à mettre en œuvre par les enseignants. Je note aussi, avec grande satisfaction, que l'obligation de l'enseignement des principes de la laïcité dans les établissements sous contrat est maintenant d'ordre législatif. alors que jusqu'à présent elle était d'ordre réglementaire et coordonnée notamment par des circulaires lesquels circulaires ne sont pas appliqués. Ainsi, un arrêté pris par le ministre de l'éducation nationale en juillet 2021 prévoit que tous les personnels enseignants de l'éducation sous contrat soient formé à la laïcité de façon obligatoire, y compris, j'insiste, ceux des établissements privés sous contrat. Or, dans les établissements sous contrat, cet arrêté aujourd'hui n'est pas appliqué. Il est même refusé d'être appliqué. J'ai été saisi, Madame la Ministre, à plusieurs reprises par des enseignants, qui regrettent l'extrême faiblesse des recrutements des formateurs dans le domaine de l'enseignement de la laïcité, ce qui est une des raisons du non-enseignement de la laïcité dans les établissements sous contrat, et ce, j'insiste, malgré les consignes du secrétariat général de l'enseignement catholique. Un certain nombre d'établissements considèrent qu'ils sont totalement libres d'enseigner ou pas la laïcité. Je pense qu'avant même l'adoption de cette proposition de loi, ce que je souhaite et j'espère qu'elle va continuer son parcours législatif, il faudrait que votre ministère s'assure de la pleine effectivité de son arrêté de juillet 2021. Merci madame la ministre, merci monsieur le président. Merci Président Ouzoulios. Nous allons examiner maintenant l'amendement numéro 1 à l'article 1er qui va être défendu par monsieur Tout à l'heure monsieur le rapporteur. Allez-y. Merci, monsieur le Président. Cet amendement porte sur l'article numéro 1. Nous trouvons effectivement très positif que la proposition de loi permette un toilettage de l'article L312-15 du Code de l'éducation qui avait enflé très largement au fil des modifications législatives de toute nature pour y inclure des sujets de préoccupation certes légitimes, nous en avons parlé, mais qui n'avaient qu'un lointain rapport avec l'enseignement moral et civique. Néanmoins, en restreignant les contours de l'EMC au strict minimum, il nous semble que certains sujets d'importance majeure pour permettre aux jeunes d'accueillir les notions essentielles à l'exercice de leur citoyenneté, sont supprimés ainsi. Il est important, nous semble-t-il, de rappeler aux jeunes que ce sont les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Il nous paraît tout aussi nécessaire de leur enseigner les principes de la République qui figurent à l'article premier de notre Constitution, soit le caractère indivisible, laïque, démocratique et social de notre République. Nous avons eu du mal un peu à comprendre le raisonnement de notre rapporteur en commission sur le rejet de ces amendements puisque les principes de la République seraient contenus dans les valeurs de la République. Et pour nous, l'indivisibilité de notre République signifie que les lois s'appliquent de la même manière pour tous. La laïcité découle de l'application de la loi 1905 de séparation des Églises et de l'État. La démocratie signifie que le peuple détient le pouvoir qu'il confie à ses représentants élus. Quant à la République sociale, ces conséquences sont multiples et impliquent un devoir de l'État pour satisfaire les besoins des citoyens en matière d'éducation, de logement et de santé. L'État est donc garant des principes de la République. Ceux-ci ne sont pas inclus dans les valeurs de liberté, égalité et fraternité. Ces valeurs obligent l'État à apporter des politiques publiques mais concernent aussi les citoyens en ce qu'ils doivent, par leur comportement et leurs actions, les respecter et les appliquer. Ainsi, l'application de l'égalité et de la fraternité implique que les citoyens ne procèdent pas à des discriminations entre eux, organisent de l'entraide ou portent des agragements associatifs. Nous sommes donc importants que l'OMC puisse éclairer les élèves sur ces deux facettes de la vie citoyenne, les principes du ressort de l'état protecteur et les valeurs partagées par toutes et par tous. Je vous remercie, monsieur le rapporteur, avis de la Commission. Oui, mon cher collègue, je reviendrai sur l'avis de la Commission qui souhaite justement l'esprit de ce texte, c'est justement de rassembler sur les valeurs de la République un enseignement moral et civique qui soit beaucoup plus concentré et qui soit moins dispersé. Et je le rappelle, pour moi, je défends les principes de la République Le groupe RDSE porte les principes et défend le principe de la laïcité, mais c'est justement parce que nous pensons qu'ils constituent les valeurs de la République, que serait la liberté sans la laïcité, que serait qu'est la fraternité, si ce n'est la solidarité, garantie justement par la laïcité des institutions, sinon ce serait du communautarisme ou du collecte. ou du corporatisme. Donc je pense qu'il est important vraiment qu'on rappelle les valeurs de la République et qu'ils sont constitués aussi des principes de la République. C'est pourquoi, pour pas à l'ourdir, on demande un retrait de cet amendement. Donc avis défavorable de la Commission. et que d'ailleurs le courrier de la Sésine du CSP mentionne bien, je cite, la transmission des valeurs fondamentales et des principes inscrits dans la Constitution. En ce titre, bien évidemment, je vous rejoins sur le fond, ce fond est déjà mentionné par écrit aujourd'hui dans nos textes. Donc c'est une demande de retrait sinon à l'avis défavorable simplement parce que je juge qu'il n'est pas forcément utile de réécrire quelque chose qui est déjà écrit. Merci. Monsieur Caner. Oui Monsieur le Président, Madame la Ministre en explication de vote. Je connais une grande élue du Nord qui dit souvent si c'est flou et vous connaissez la suite. Monsieur le rapporteur, madame la ministre, je ne sais pas pourquoi les explications qui ont été données par notre collègue Adelzian, permettant finalement de préciser l'esprit et la pratique pour l'EMC, autour notamment des valeurs de laïcité, ne pourraient pas apparaître en tant que tel dans la loi. Il y a eu une simplification à tous les tâches d'une chose, Mais il ne faudrait pas que le toilettage aboutisse finalement à réduire à portions congrues ce qui fait notre pacte républicain, notre promesse républicaine et notre vivre ensemble. Donc nous, nous pensons qu'il faut inscrire dans la loi, dans le texte proposé par monsieur Cabanel, ces éléments complémentaires. Je ne sais pas de quoi vous avez peur. C'est net, c'est clair. Il faut montrer notre engagement. Et je me souviens de propositions, et en l'occurrence même de projets de loi du gouvernement, visant à ce que la question de la laïcité soit parfaitement identifiée, y compris dans les relations entre l'État et les associations. Eh bien, nous, nous allons dans ce même sens, Madame la Ministre.

Je ne sais qui c'est qui a levé le doigt en premier, mais monsieur Zoulias... Merci monsieur le Président, madame la Ministre, mes chers collègues, Jean Raymond Hugonet, je crois qu'on va avoir le même discours, donc vous me conforterez, et je voulais vous citer prioritairement, parce que pendant le temps que vous avez passé à la Commission de la Culture, vous nous avez instruit sur la différence essentielle entre valeur de la République et principe. Vous me permettrez d'en... revenir au latin mais la valeur c'est ce qui vaut, c'est-à-dire c'est ce qui se mesure. Les principes c'est ce qui est premier. Et c'est quelque chose de totalement différent. Et je pense que dans un texte de loi comme celui-là, faire référence à l'article premier de la Constitution, ça me semble vraiment une évidence. Je ne comprends pas votre opposition. La Constitution, c'est la loi commune. Faire référence quand on s'adresse aux élèves, ça me semble une absolue différence. Cher collègue Gonnet, je vous laisse le soin de compléter mon analyse. mais j'ai déjà emprunté un certain nombre de vos arguments et je m'en excuse. Merci M. le Président. Donc, comme il vous l'a suggéré, à vous, M. Huygonet. Merci. Merci M. le Président. Je dois vous dire que je suis assez heureux de ce débat, ce matin, parce que voilà six ans, depuis que je suis rentré dans cette maison, que je me bats pour que le distinguo subtil, mais pourtant évident, entre les valeurs de la République qui sont très claires, qui sont au nombre de trois et que tout le monde en France, je l'espère encore, connaît, liberté, égalité, fraternité, mais que les principes de la République sont également énoncés dans ce document qu'on a tous oublié, sauf ici, je l'espère, qui s'appelle la Constitution de 1958 et la laïcité est un principe. Pendant six ans, j'ai repris deux fois, deux fois, les deux ministres successifs de l'Éducation nationale qui commettaient Alors, comment dire ? Je ne veux pas dire par incompétence, je ne me permettrai pas. Et si c'était pas de l'incompétence, c'était Siaman qui mélangeait les valeurs et les principes. Et ils n'étaient pas à l'aise quand on leur posait la question, quand je leur posais la question lors des auditions, parce que tout simplement, c'est faire une erreur fondamentale. Bien entendu, notre pays est laïque. Nous en sommes fiers. On a même inventé cette laïcité. En revanche, Il ne faut rien toucher à ce qui existe, qui est clair, qui respecte tout le monde. Les valeurs de la République sont très claires, les principes en font partie, mais les valeurs sont premières. Et merci à Pierre Ouzoulias d'avoir rappelé ces débats aux mairies et aux présidents Lafond qui est au banc. Merci beaucoup, cher collègue. La parole est maintenant à monsieur Cabanel qui l'avait demandé. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. J'ai bien entendu ce qui vient d'être dit, et en tant qu'auteur de la proposition de loi, je le pense et je suis assez favorable à ce qui vient d'être dit. Je crois qu'il est important de penser laïcité, mais de le dire, c'est encore mieux. Donc je voterai cet amendement. Merci, oui. Le monde va mal et lorsque l'on parcourt ce monde et lorsque ceux d'ailleurs nous parlent de la France et de son patrimoine, on nous parle évidemment des objets patrimoniaux de notre pays. Mais quand on parle du patrimoine immatériel de la France, on nous parle évidemment de ces grands principes de la République et notamment de la laïcité. Vous savez, les valeurs, lorsque vous écoutez dans cet hémicycle ou ailleurs, quel que soit le bord, on peut interpréter les valeurs à sa façon. Et chacun, d'ailleurs, réinterprète la notion de valeur à sa façon. Mais les principes, eux, sont intangibles. Et si nous avons quelque chose d'exceptionnel à faire valoir dans ce monde qui va mal et dans notre pays, c'est bien la laïcité. Et c'est à la laïcité qu'il faut se référer et à ces principes. Et quand un principe est bien énoncé, eh bien, il s'entend mieux. Voilà. Je soutiendrai cet amendement. Merci, cher collègue. Madame la Ministre, je crois que vous vouliez la parole. Merci, Monsieur le Président. De façon à très clair, bien évidemment, nous devons en permanence rappeler les valeurs et les et les principes de notre République. Et ce n'est pas en tant que secrétaire d'État en charge de l'engagement du SNU et de la vie associative que je dirais le contraire. Simplement rappeler que déjà aujourd'hui, dans nos textes, les valeurs, les principes de notre République sont déjà inscrits, que le respect qu'il se doit de façon extrêmement stricte est déjà inscrit et consigné, et que, selon moi, il ne s'agit pas de venir écrire à nouveau ce qui est déjà écrit, mais bien, et je vous rejoins, M. le Sénateur, de faire appliquer strictement ce qui, justement, est écrit. Et c'est justement cela qui péchait avant. Parce que, effectivement, jusque-là, il y avait effectivement un flou. Et quand il y a un flou, je vous rejoins parfaitement. Et c'est la raison pour laquelle le ministre... Je vais finir juste mon propos. Laissez-moi finir mon propos, vous allez voir, ça va être peut-être plus clair. Et justement, l'enjeu qui a été celui de Gabriel Attal dès sa nomination au sein de l'Éducation nationale et de la jeunesse, ça a été de sortir des zones grises sur l'ensemble des sujets que vous venez de mentionner. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est justement bien appliquer l'enjeu que nous avons de faire en sorte. Ce n'est pas de se dire est-ce que nous sommes d'accord sur les principes et les valeurs de notre République ici. Je pense que nous le sommes. C'est de faire en sorte que ce soit appliqué à l'extérieur de cette enceinte justement. Merci. Merci. Je vais donc mettre au voix cet amendement numéro 1 qui a reçu un double avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Que ceux qui souhaitent l'adopter le fassent en levant la main. Qui est pour Qui est contre ? Qui s'abstient ?

Merci Président. Dans le même ordre d'esprit, effectivement, le travail de toilettage qui est effectué dans le cadre de ce projet de loi pour resserrer les contours de l'EMC. Évidemment, nous l'avons évoqué précédemment, faire porter sur cet enseignement tous les sujets de préoccupation légitimes n'ayant qu'un lointain rapport avec la formation d'une citoyenneté responsable n'est ni raisonnable ni réaliste et nous partageons ce constat. J'en veux pour preuve les objectifs qui figurent actuellement à l'article L315 du Code de l'éducation, sensibilisation à la maltraitance animale, mise en garde contre les produits fabriqués par des enfants, etc. Et j'en passe. On se demande d'ailleurs quand, et nous l'avons évoqué, les professeurs des écoles ou d'histoire géographique trouveraient le temps d'aborder la diversité de ce sujet dans le cadre de l'EMC, notamment à raison d'une heure en primaire et d'une heure toutes les deux semaines au lycée. Néanmoins, nous voulions alerter là-dessus, on ne peut pas rayer d'un trait certains sujets qui s'inscrivent parfaitement dans le cadre d'un apprentissage à la citoyenneté qui doit demeurer l'objectif de l'EMC. Ainsi, nous souhaitons que demeure du ressort de l'EMC la sensibilisation des élèves aux dangers de l'Internet et à la manipulation de l'information, ainsi qu'aux droits et devoirs des enfants et à toute forme de maltraitance et de harcèlement les concernant, en particulier à l'heure où le ministre de l'Éducation a décrété grande cause la lutte contre le harcèlement scolaire. L'apprentissage de ces notions est essentiel à la formation de citoyens, libres, égaux et fraternels. Notre rapporteur nous avait indiqué en commission que ces atouts seraient redondants avec des dispositifs de code de l'éducation qui ont déjà inscrit qui ont déjà inscrit des objectifs de l'enseignement scolaire. Un article liminaire du code de l'éducation affirme en effet qu'aucun élève ne doit subir de harcèlement, mais affirmer un principe est positif, mais cela n'inclut pas qu'un enseignement sur le sujet soit dispensé. Quant aux exigences de sensibilisation à la manipulation de l'information ou d'information sur le droit des enfants, elles ne figurent aujourd'hui qu'au titre des anciennements dispensés lors de l'EMC, dispositif que cet article supprime. J'estime très lourd ces conséquences et c'est pourquoi nous souhaiterions que ces sujets restent de la compétence de l'EMC et soient gravés dans la loi. Avis de la Commission. Monsieur le rapporteur. C'est jusqu'à preuve du contraire, encore un avis défavorable, parce que le ministre que nous avons auditionné il n'y a pas très longtemps nous a dit d'ailleurs qu'il voulait faire de l'EMI, justement qui ne rentrera pas dans l'EMC, mais l'EMI aussi une des priorités des programmes de l'enseignement et je pense qu'il faut donc appeler un chat un chat, il y a l'enseignement moral, civique, qui doit revenir sur les valeurs et maintenant les principes de la République, et ensuite l'enseignement sur les médias et l'information avec tous les risques que vous avez cités, avec toute l'importance qu'elle revêt et que nous défendons, qui doit entrer dans un autre programme qui est celui de l'OMI, qui a été très clairement ciblé par le ministre de l'éducation nationale. C'est pour cette raison que nous avons donné un avis défavorable à cet amendement. Merci monsieur le rapporteur, madame la ministre, pour le gouvernement. Merci Monsieur le Président, à nouveau si je vous rejoins sur le fond, c'est sur la forme que nous allons avoir une différence, parce que vous le dites de façon très juste, c'est qu'aujourd'hui le risque c'est de demander tout à l'EMC au risque qu'il ne soit plus assuré la complétude. de ce temps d'enseignement extrêmement important au regard du texte que nous sommes aujourd'hui en train de débattre. Cela a été rappelé aussi bien par le rapporteur et déployé par le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, Gabriel Attal, le déploiement de l'attestation PIX qui est déjà prévue d'ailleurs sur toute la scolarité de la troisième à la terminale dans cet esprit justement de développer cette capacité à se saisir aujourd'hui des outils numériques pour les encadrer, les structurer et lutter aussi contre le fléau que nous dénonçons et sur lequel nous devons achir collectivement qui est le harcèlement et donc le cyber cyber harcèlement également. Donc encore une fois ce n'est pas en enjeu d'être contre votre amendement puisque il est satisfait et il est d'autant plus satisfait qu'aujourd'hui il est aussi traité sur un temps particulier, à part entière, qui assure sa pleine complétude dans le cadre des enseignements de nos enfants. Donc c'est donc une demande de retrait, sinon un avis défavorable. la ministre, a demandé la parole. Oui, simplement pour rajouter ce que vient de dire le rapporteur et madame la ministre. Monsieur Zian, vous êtes maintenant avec nous à la Commission depuis quelques semaines. Vous l'avez entendu, bien évidemment dans l'absolu, il faudrait que dans le cadre de l'école, on puisse parler au-delà du harcèlement. du respect du corps, de la sensibilisation à la sexualité dès le plus jeune âge. Je vois Mme Monnier qui est à côté de moi et qui en a fait aussi un combat comme nous. Et on ne peut pas mettre tout ça dans le peu d'heure qui est accordé à l'EMC. Il faut bien évidemment pouvoir en parler à l'école, mais c'est vrai que si on pouvait se recentrer comme l'a fait l'auteur du texte et le rapporteur sur vraiment la citoyenneté et la valeur de la République, C'est important. Mais j'espère qu'en effet, Madame la Ministre, ces différents sujets qui sont primordiaux, parce qu'on voit des atteintes notamment, comment dire, atteintes à la sexualité aux victimes dès le plus jeune âge, il faut bien évidemment qu'on puisse en parler dans le cadre de l'école.

qui est contre, qui s'abstient, il n'est pas adopté. Je vais mettre au voie maintenant l'article premier qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté.

Mes chers collègues, si le régime du Concordat prévoit l'existence d'un enseignement religieux à l'école publique dans les départements du Bahrein, du Horrain, de la Moselle, une faculté de dispense est néanmoins prévue pour les familles qui souhaitaient dispenser les élèves de cet enseignement. Dans le premier degré, cette dispense est formalisée à l'article D 481-6 du Code de l'éducation, qui prévoit que les enfants dispensés de l'enseignement religieux réglementaire reçoivent au lieu et place de l'enseignement religieux un complément d'enseignement moral. Dans le second degré, cette dispense est organisée par voie réglementaire. Or, s'il est prévu dans les textes, cet enseignement moral n'est pas effectif dans la pratique. Les parents d'élèves de ces départements témoignent ainsi que les élèves qui ne suivent pas l'enseignement religieux ne se voient pas délivrer de contenus pédagogiques pendant cette heure de dispense, les réduisant à de l'occupationnelle. Quelques exemples d'activités parmi celles qui m'ont été remontées, coloriage, dessin libre, lecture libre. Cela conduit mécaniquement à une perte de 180 heures d'enseignement obligatoire pour les élèves concernés. Devenus majoritaires en Alsace comme en Moselle, le taux de participation à l'enseignement religieux serait en effet passé en dessous de 50% pour l'école primaire. Nous ne pouvons que déplorer cette situation d'autant plus au cours de l'examen d'une proposition de loi qui insiste sur le rôle socle que doit jouer l'enseignement moral civique dans l'éducation citoyenne de nos élèves. Afin de faire la pleine lumière sur ce sujet, cette amende m'envise par conséquent à demander la remise de rapport sur l'effectivité de l'organisation de l'enseignement moral complémentaire auxquels les élèves des établissements du premier degré dispensés d'enseignement religieux dans les départements du Bahrain, du Haut-Rhin et de la Moselle doivent être soumis qui proposeraient le cas échéant des pistes pour rendre plus effectif cet enseignement complémentaire. Je vous remercie. Un vie de la Commission. Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président. Oui, mes chers collègues, vous connaissez la coutume du Sénat qui est de refuser les rapports. En revanche, et ce n'est pas M. Ousoulias qui me démentira, c'est un sujet qui peut nous intéresser et je m'étais engagé à demander donc au gouvernement Puisque nous ne demandons pas de rapport, au moins d'avoir une information, cette information sur cet enseignement qui doit se substituer à l'enseignement religieux en Alsace et Moselle comme l'impose la loi. Donc avis défavorable et attente de cette information par le gouvernement. Merci, avis du gouvernement, Madame la Ministre. Même avis, donc. Je vais... Monsieur Ousoulias, Président Ousoulias. Merci Monsieur le Président. Madame l'Alliche, chers collègues, votre défense est un peu courte. J'aimerais rappeler que l'enseignement de la religion, Alsace-Moselle est imposée par une loi allemande du 10 juillet 1873. Ça n'a rien à voir avec le concordat. Il faut bien distinguer le droit local et le concordat. Je le répète, cette loi allemande imposée par le Reich au département occupé, demande d'enseigner la religion. Ce qui est très différent de l'enseignement sur les religions, tel qu'on l'a dans les établissements publics de la France de l'intérieur, pour parler comme les Alsaciens. Ce que je retiens des chiffres de fréquentation de 2022, mais malheureusement le ministère ne nous a pas communiqué des chiffres plus récents, c'est qu'en Moselle, cet enseignement de la religion est suivi par 35% des élèves pour le primaire, au collège c'est 7% et au lycée c'est Pour l'Alsace, la part de fréquentation de ces cours au lycée est de 20%. Donc nous sommes dans le cas tout à fait particulier d'un enseignement qui est obligatoire et pour lequel les dispenses d'enseignement sont majoritaires. ce qui pose quand même un problème. Je pense qu'il faudrait que le ministère se pose la question si, alors je sais que c'est très difficile de toucher au droit local allemand mais là en l'occurrence on pourrait peut-être rapprocher l'enseignement de la religion de l'enseignement des faits religieux tels qu'il est pratiqué dans les autres établissements et je vous conseille de de relire l'excellent rapport de Régis Debray sur le cas qui montrait la nécessité justement d'enseigner les religions, c'est-à-dire d'une forme de distanciation critique par rapport à la religion elle-même. Je remercie monsieur le Président. Merci, la parole est à madame Monnier. Oui madame la ministre, je souhaiterais que vous apportiez une réponse parce que d'abord monsieur le rapporteur a été très clair et vous a redonné et on est tous en fait en train de dire qu'on ne peut pas laisser les choses en état et qu'il faut savoir où on en est et ce qui est fait. Vous madame la ministre ? Effectivement. En fait, ce que je peux vous proposer, c'est d'organiser une mission d'inspection générale sur le sujet. Ça va d'autant plus loin que ce qui est proposé et ce qui est demandé, si cela vous va, bien évidemment, et on pourrait faire effectivement un état des lieux sur la mise en œuvre en complémentarité, en subsidiarité, comme vous venez de le dire, si cela vous va. Je mets donc au voie cet amendement avec un double avis défavorable du gouvernement et de la Commission, Qui est pour ? Qui est contre ? Et qui s'abstient ? Il n'est pas adopté. Article 2, amendement numéro 3. Monsieur Zien. Merci Président. Cet amendement vise à réintroduire dans le dispositif de l'article du Code du service national qui définit les modules dispensés lors de la Journée de défense citoyenneté des exigences qui sont dans l'esprit que nous sommes en train d'étudier ce matin de rationalisation, de toilettage, de nettoyager un petit peu des thématiques. Il nous semble dangereux aussi à un certain moment, enfin dommageable, qu'un certain nombre de thématiques soient exclus. Et ces exigences portent justement sur des thématiques portant sur le respect de l'égalité des sexes doit être un moteur important de l'intégration des femmes dans les armées, surtout à l'heure où les femmes représentent près de 17% des effectifs de l'armée française et que plus aucun poste ne leur est interdit. Il nous semble aussi important que cette journée axée sur les possibilités d'engagement dans les forces armées et de réserve ne soit pas un moment d'autocensure pour les femmes pour postuler dans les armées et nous souhaitons que ces éléments puissent réintégrer. De formation également puisqu'elles disparaissent, ces éléments disparaissent de formation sur la lutte contre les préjugés sexistes ou homophobes. Même critique que celle émise précédemment également sur les autartiques puisque comme pour les femmes, toutes les personnes également homosexuelles doivent être pleinement intégrées dans ce corps qui leur a encore jugé hostile. Et enfin, un autre élément qui disparaît des éléments de réflexion et d'apprentissage au cours de cette journée, la formation contre les violences conjugales et commises au sein du couple. Pour nous, enfin, les formations qui doivent être dispensées doivent permettre de sensibiliser ces derniers, que ce soit dans le corps militaire, en faisant des relais de ces causes dans tous les organes possibles. Je vous remercie. Oui, monsieur le Président, donc mes chers collègues, c'est sûr que Oui, monsieur le Président, donc mes chers collègues, c'est sûr que l'égalité homme-femme, la lutte contre l'homophobie, les préjugés sexistes, l'information sur les violences faites au sein des couples, c'est vraiment des sujets très importants. En revanche, est-ce qu'ils ont vraiment leur place dans la journée défense citoyenne où justement l'objet donc de cette proposition de loi c'est de ramener sur l'essentiel de l'information qui doit passer sur la défense et la citoyenneté Et c'est des sujets qui, on l'espère, doivent être traités, et il faut veiller tout au cours de la scolarité et de la formation des citoyens, mais qu'on revienne justement l'esprit de cette proposition de loi, c'est de revenir à l'essentiel et aux informations, et entre autres que cette journée de défense citoyenne laisse une place plus importante que les trois heures actuelles sur les informations, sur la défense, sur les métiers qui sont proposés, d'ailleurs aux femmes comme aux hommes, sans préjuger d'ailleurs des orientations sexuelles des gens qui vont y participer. Donc un avis défavorable de la Commission. Madame la Ministre, pour le gouvernement, même avis. Je vais mettre au voie l'amendement n°3 qui a reçu un double avis défavorable de la Commission et du gouvernement, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il n'est pas adopté. Je vais maintenant mettre au voie l'article 2 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il est adopté. Article 3, amendement du rapporteur, amendement n°5, pour lequel je pense bien évidemment qu'il sera favorable. cet amendement est là pour rassurer d'abord le gouvernement et fait suite d'ailleurs à une remarque en audition du président Stéphane Piednoir qui pouvait s'inquiéter sur le fait de prolonger de trois à six mois la possibilité de garder dans les épides des jeunes qui, suite à un emploi ou un stage n'aurait pas d'hébergement, eh bien c'est donc de dire que ce renouvellement de trois mois supplémentaires se ferait en fonction, dans la limite, des places disponibles. Je rappelle qu'il doit y avoir à peu près entre 5 et 10% des places qui le sont. qu'un grand progrès avait d'ailleurs été fait puisqu'au début les jeunes qui étaient dans les épides n'étaient pas hébergés le week-end et qu'on voyait des jeunes qui retournaient parfois coucher dans la rue pendant les week-ends et revenaient ensuite. Donc ça a été élargi puisque maintenant ils peuvent rester dans les week-ends et là c'est de leur permettre de rester trois mois supplémentaires s'ils n'ont pas de solution d'hébergement. Ça fait partie, je crois, du du parcours nécessaire pour ces jeunes. Merci monsieur le rapporteur, madame la ministre. En toute logique c'est un avis favorable bien évidemment et monsieur le Président si vous me le permettez est en lien étroit avec le texte que nous étudions aujourd'hui qui va justement sur le sujet de la citoyenneté, de faire vivre la citoyenneté au quotidien de façon très claire pour l'entièreté de nos jeunes et moins jeunes d'ailleurs aussi. avec cette nécessité d'être dans l'inclusion et de la connaissance de nos institutions institutions aussi bien locales, nationales qu'européennes. Je tiens aujourd'hui à saluer Thomas, qui m'accompagne aujourd'hui dans le cadre du DOD et qui va aujourd'hui donc découvrir le fonctionnement du Sénat dans l'intéreté de son Sénat et de cette institution et qui me suivra cet après-midi à Bruxelles. Je vous remercie pour son accueil aujourd'hui. Merci. Monsieur Ziane. Petite réaction rapide aux explications de vote. Effectivement, ça a été évoqué. Le taux d'occupation d'occupation moyen dans les épides est actuellement compris entre 90 et 95 %. Et cet amendement précise que le revenement trois mois de l'hébergement se fait dans la limite des places disponibles. Nous interrogeons un petit peu parce que nous trouvons que c'est réducteur par rapport à l'ambition du dispositif initial qui donnait droit à tout volontaire pour l'insertion, apprenti ou en contrat temporaire ou en contrat de professionnalisation, lorsqu'il a trouvé un emploi avant la fin de ce contrat, de bénéficier pendant trois mois des prestations, des pides dont un logement. Il nous semble très clairement qu'à travers cet amendement cette possibilité est réduite dans la limite donc des places de logements disponibles. Il n'y aurait donc aucune obligation de maintenir cette possibilité de logement aux jeunes et je comprends la problématique des moyens et des objectifs mais si le parc est occupé à 90-95% comme mentionné dans l'objet, le dispositif devient donc juste une déclaration de principe et ne sera pas utile. Je vous remercie, ils nous ils nous abstiendront. Merci, je vais donc mettre au voie Cet amendement numéro 5 a reçu un double avis favorable de la Commission, bien évidemment, puisqu'elle en est l'auteur, et du gouvernement qui est pour, qui est contre, et qui s'abstient. Il est adopté. Article 3, j'imagine le même vote, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, est adopté. L'article 4 que je vais mettre au voie, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il est adopté. Madame, je suis saisie d'une demande de parole de Madame la Présidente Cécile Cuckerman. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Je veux, à travers cette prise de parole, je crois attirer l'attention et je ne fais pas bien évidemment offense à nos collègues dans la rédaction de cet article 5 sur ce qui pourrait apparaître demain être une fausse bonne idée et qui serait l'accélération de la dématérialisation de l'envoi de la propagande électorale. nous avons déjà dit, nous avons eu d'autres textes, nous sommes dans une crise politique, dans une crise de confiance. Tout d'abord, je veux rappeler ici avec solennité que l'envoi de la propagande électorale ne peut être assimilé à tout autre prospectus de réclame ou d'autres choses qui peuvent fleurir dans les boîtes aux lettres. Je crois que nous devons nous préserver parce que même si nous allons vers simplement une démarche volontariste, il pourrait y avoir un écueil d'un certain nombre de nos concitoyens qui, parce qu'ils ne veulent plus entendre parler de tout ça, cocherait de manière un peu rapide la dématérialisation de l'envoi de la propagande électorale pour finalement ne plus avoir et regarder de plus près. Donc je crois que c'est quelque chose que nous devons manier avec vraiment j'ai eu à d'autres occasions ici dans ce semicycle l'occasion de le dire je crois que c'est l'exercice de la propagande électorale de la de la profession de foi et du bulletin de vote qui est finalement le dernier rapport qu'a les lecteurs à la veille de son scrutin avec son choix à faire demeure importante et je voudrais d'ailleurs rappeler au combien et nous avons d'ailleurs parfois même été surpris les uns et les autres de l'émotion de 2021 quand au moment des élections départementales et régionales, une grande partie de nos concitoyens n'ont pu recevoir ce matériel électoral pour les différents problématiques que d'ailleurs le président Buffet dans la commission de contrôle qui en avait suivi avait démontré. nous ne nous opposerons pas à cet article 5, mais je veux le dire, ne généralisons pas trop vite Ces dématérialisations qui pourraient demain être des fausses bonnes idées dans le rapport de nos concitoyens avec les choix électoraux et donc les choix civiques. Merci Madame la Présidente. Je vais mettre au voie l'article 5 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il est adopté. Je mets au voie maintenant l'article 6 qui est pour. qui est contre, qui s'abstient, est adopté. Je mets au vote l'article 7, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Je vais mettre au vote l'ensemble de la proposition de loi. Y a-t-il des demandes d'explication de vote ? Je n'envoie pas. Monsieur l'auteur de la proposition de loi, Henri Cabenel. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Comme j'ai pu le dire dans mes propos liminaires et comme ça a été dit et partagé sur tous les bancs, cette proposition de loi n'est certes pas très ambitieuse, mais elle est l'objet donc d'un compromis puisque, sur certains points, dans ces bannes de l'hémicycle, nous ne sommes pas tout à fait en phase. Donc, je pense qu'il faut, pour aller loin, aller doucement. Et dans le cadre donc de cette proposition de loi, ce qui a été et qui me semble être partagé par tous, ce sera déjà un premier pas. Je ne comprends pas tout à fait les arguments que vous développez, Madame la Ministre, sur les articles dont vous n'êtes pas d'accord et notamment sur un qui me semble essentiel, c'est le statut de l'étudiant élu. Parce qu'aujourd'hui, dans la Convention nationale des élus locaux que votre gouvernement a engagé, à travers la ministre Dominique Faure, c'est une volonté des élus locaux d'avoir un véritable statut. Là, on consacre cette PPL vers les jeunes, où on se tousse, on fait le constat que ce sont eux qui se déplacent le moins quand même aux élections, et pour favoriser justement leur engagement, on crée un statut. Je pense que ça serait un mauvais signe de votre part que de rester dans cette attitude-là, parce que je crois que c'est une demande forte des jeunes qu'on a pu rencontrer, parce que Moi, si je dois retenir quelque chose de la mission, c'est qu'à travers toutes les auditions que l'on a pu faire, j'ai souhaité à un moment donné qu'on fasse la place aux jeunes. Et on a écouté les jeunes. Et les jeunes, eux, c'est un besoin pour eux. Et donc, voilà, je voulais le signifier. En tout cas, je tiens à remercier tous mes collègues qui apparemment sont d'accord sur cette proposition de loi. Bien sûr, la Commission culture et son rapporteur Bernard Fialer. En tout cas, c'est une avancée et je suis, comme vous, persuadé qu'il va falloir aller plus loin, mais il va falloir le faire toujours dans un compromis pour pouvoir avancer. Merci. Merci. Alors Alors si nous voulons examiner la prochaine proposition de loi, je vous demande d'être rapide, monsieur Jeanne, vous avez demandé la parole, Merci président, pour quelques mots, remercie aussi le travail qui a été effectué en commission, les échanges respectueux que nous avons pu tenir les uns avec les autres. Trois points, évidemment, notre souhait dans ces débats, il était essentiel pour nous qu'un certain nombre de thématiques qui nous semblaient disparaître de l'EMC ne soient pas renvoyées vers d'autres dispositifs dont les contours ne sont pas encore clairs, dont les contours ne sont pas forcément tous et tous bien étayés et bien considérés. Le deuxième point, sur la question des principes et de la dissection entre les principes et les valeurs de notre République, C'est un sujet qui nous tenait particulièrement à cœur et je remercie aussi l'ensemble des collègues d'avoir pu en débattre sereinement. Et enfin, troisième point, sur ce statut de l'étudiant, je remercie encore le sénateur Cabanel de cette mission et des informations et des propositions qui ont été déposées, fait écho aussi au Congrès des maires qui s'est tenu, qui se tient actuellement, des discussions qui ont pu avoir lieu au sein des enceintes diverses et variées. Et ce point-là, il faut être en capacité de proposer à des étudiants qui souhaitent s'engager aujourd'hui et proposer une véritable envie de se porter dans l'engagement politique des citoyens, de leur proposer un statut qui, à l'âge dans lequel ils sont, entraîne des difficultés parfois particulières en termes de financement, de capacité à financer cet engagement politique. Je vous remercie. J'espère conclure avant que nous passions au vote. au vote. Très rapidement et pour répondre effectivement sur le sujet du jeune étudiant effectivement et des étudiants et des jeunes qui sont effectivement élus, oui on en a parlé et je vous rejoins, je suis complètement d'accord sur ce principe-là. Le texte est dans son début de travail législatif et de véhicule C'est un sujet qui importe de travailler en plus profonde adéquation avec le Ministère de l'Intérieur. Je serai absolument ravie de me tenir à votre disposition pour que nous puissions avancer dans ce cadre-là, dans la suite du véhicule législatif. Voilà, je vais donc mettre au voie l'ensemble de la proposition de loi tendante à renforcer la culture citoyenne qui est pour qui est contre, qui s'abstient, celle-ci est adoptée. Alors je vais suspendre la séance quelques instants afin de permettre à chacun de s'installer pour le prochain point à l'ordre du jour. La séance est suspendue.

Cher collègue, l'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi visant à aménager la prévention des risques liés au bruit et au son amplifiés, présenté par Madame Nathalie Delattre et plusieurs de ses collègues demande du groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Dans la discussion générale, la parole est à l'auteur de la proposition de loi, Madame Nathalie Delattre, pour dix minutes. Merci M. le Président, Mme la Ministre, M. le Président de la Commission, M. le Rapporteur, mes chers collègues. L'entrée en vigueur du décret du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés au bruit et au son amplifié, dit décret bruit, a modifié l'article R13366 du Code de la santé publique. Cette modification, qui trouve son origine dans la loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé, a fait basculer l'ensemble des activités de sport mécanique dans le droit commun des bruits de voisinage. Cette évolution soumet de fait les sports mécaniques à un dispositif d'infraction pénale, plaçant de très nombreux circuits et surtout la pratique encadrée de ces sports dans l'incapacité de respecter la règle d'émergence. Elle porte en germe des risques contentieux bien réels qui menacent la pérennité des activités sportives des fédérations françaises de sport automobile et de motocyclisme. En effet, aucun circuit ne peut raisonnablement respecter ce nouveau cadre réglementaire disproportionné. Un cadre qui a malheureusement fait fi de la situation des sports mécaniques puisque ces acteurs n'ont à aucun moment été associés aux discussions préalables à la mise en œuvre de ce décret d'application. Par cette proposition de loi, il s'agit de trouver une solution équilibrée, partageant l'objectif ciblé et pragmatique de création d'un régime proportionné contre le bruit conciliant pratique des sports mécaniques et protection de la tranquillité publique. À aucun moment l'objet de cette proposition de loi n'est d'autoriser un bruit accessible et nuisible à la santé. Les circuits de sport mécanique font partie du patrimoine collectif de notre pays. Environ 2 300 épreuves sportives sont organisées chaque année à travers notre territoire sur plus de 1000 circuits, dont 37 circuits de vitesse. Ils sont le porte-étendard du savoir-faire français en matière de sport mécanique, où l'aura et la popularité auprès d'un public varié des compétitions, tels que les 24 heures du Mans ou le Grand Prix de France de Formule 1, dépassent largement nos frontières hexagonales. Je rappelle que la filière des sports mécaniques en France est aujourd'hui 2,3 milliards d'euros annuels d'impact économique et 13 500 emplois directs, la propulsion troisième filière économique et sportive en France. Autour de chaque site, c'est tout un écosystème générant des emplois directs et indirects qui s'est tissé, un fermement de cohésion sociale et d'animation de nombreux territoires tant ruraux qu'urbains. Cette épée de Damoclès qui pèse ainsi sur la continuité de ces activités ne peut perdurer et une solution aménageant les contraintes qui pèsent tant sur les fédérations de sport mécanique que sur les acteurs des circuits automobiles tout en garantissant le respect des normes de sécurité et de protection de l'environnement doit être trouvée. Aujourd'hui, les fédérations sportives délégataires doivent se conformer à une réglementation complexe, rendant l'application de ce décret bruit d'autant plus excessive. Après l'obtention d'un arrêté d'homologation de la part du préfet, qui se renouvelle tous les quatre ans, après visite et avis de la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse ou de la Commission départementale de sécurité routière, elles édictent dans le cadre de leur mission de service public les règles techniques et de sécurité dont les réglementations sonores font déjà partie intégrante. Désormais, dans l'impossibilité de respecter la règle d'émergence prévue par le nouveau cadre juridique en vigueur, identique à celle des activités industrielles, ne relevant pas du régime ICPE, c'est-à-dire inférieur à 5 décibels en journée et 3 décibels en période nocturne, de nombreux circuits se trouvent à portée de fermeture d'une seule plainte émanant d'un riverain ou d'un collectif. Une menace qui se renforce à mesure que l'urbanisation se déploie et s'étend à proximité des circuits pourtant initialement construits en périphérie des centres urbains pour ne pas être une gêne. D'autant que l'article L113-8 du Code de la construction et de l'habitation, qui prévoit l'opposabilité de l'antériorité de la construction aux activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, ne s'applique pas aux sports mécaniques. Cette menace est d'autant plus paradoxale que la filière des sports mécaniques est vectrice et propice aux innovations technologiques et techniques en matière environnementale. La France est pionnière en la matière avec une réduction de plus de 20 décibels en 20 ans des émissions sonores à la source des véhicules. Reconnue pour ses compétences et son excellence dans le domaine de l'ingénierie automobile, de la conception des moteurs aux pneumatiques, la filière a développé de manière significative, par le biais de ses fédérations et constructeurs, de nouvelles technologies profitant à l'ensemble de l'industrie automobile, à l'ensemble des citoyens que nous sommes. À l'origine de la motorisation hybride ou électrique et du biocarburant, les compétitions de sport mécanique catalisent et transposent les avancées technologiques et techniques réalisées sur ce circuit vers nos véhicules de série. Entraver leur développement, c'est par conséquent ralentir l'indispensable transition écologique des transports qui, je le rappelle, reste la première source de gaz à effet de serre sur notre territoire. Du reste, comme preuve de leur volonté de poursuivre leurs efforts en la matière, la Fédération française du sport automobile et la Fédération française de motocyclisme seront les deux premières fédérations françaises sportives à rendre, et ce sera au début du mois de décembre prochain, les conclusions du baromètre environnemental qu'elles viennent de mettre en place. Par ailleurs, ne pas agir devant le risque de paralysie de l'économie des sports mécaniques, c'est aussi prendre le risque que se développent les rodéos urbains. Dois-je vous rappeler qu'il y a 50 ans, le gouvernement avait justement décidé le développement de nombreux circuits de sports mécaniques afin de répondre aux problématiques de rodéos urbains et à leurs conséquences tragiques. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le circuit situé à Tremblay en France s'appelle le circuit Carole, prénom de la dernière victime déplorée avant la création du circuit. Il ne s'est en outre jamais autant vendu de motos ces dernières années. N'est-il pas préférable d'encourager une pratique encadrée sur circuit que de voir ces derniers fermer un à un, menant inéluctablement au développement de ces rodéos urbains ? Et je suis bien placée en Gironde pour en attester. De nombreux maires m'ont fait part de leur soutien à l'occasion de ma PPL, et je salue madame le maire Dalhuy dans les tribunes, faisant le souhait de ne pas perdre leur circuit dans leur département. Ils ne veulent pas voir se développer la conduite hors cadre, qui d'ailleurs, comble de la situation, ne serait soumise à aucune mesure de bruit puisque la voie république bordée de millions d'habitations n'est pas concernée par ce décret bruit. C'est donc, chers collègues, dans toutes les raisons que je viens d'évoquer, que cette proposition de loi trouve son essence. Elle ne crée pas un droit à la pollution sonore. Elle ne propose pas de retour en arrière, ni un blanc-sain au sport mécanique pour faire du bruit. Elle propose de trouver un compromis entre survie des circuits et et santé publique. Et ce compromis se matérieuse lise par l'introduction d'une dérogation à l'article L567116 du Code de l'environnement. Ce dernier prévoit initialement que les activités bruyantes sportives et de plein air ainsi que les activités bruyantes exercées dans les entreprises, les établissements et les centres d'activité où les installations publiques ou privées établies à titre permanent ou temporaire et ne figurant pas à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement peuvent être soumises à des prescriptions générales voire à une procédure d'autorisation. La dérogation serait ainsi applicable au seul sport mécanique, prévoyant qu'il soit soumis à ses dispositions particulières, précisé par décret, tenant compte des contraintes propres à leurs activités. Cette loi permettrait ainsi au pouvoir réglementaire de modifier le décret bruit de 2017 et d'accompagner la transition technologique et technique des acteurs des sports mécaniques, plutôt que de continuer à imposer des normes inapplicables, car disproportionnées. à plonger cette filière dans le marasme et la sécurité routière en grand danger. Enfin, je souhaite remercier le rapporteur Alain Dufour et son administrateur pour leur travail très consensueux et positif et mon groupe d'avoir inscrit ce texte à son ordre du jour. Il nous incombe à présent, chers collègues, de débattre en conscience et dans le temps. J'aimerais effectivement que ce texte puisse être voté avant 13h, sinon nous serions obligés de l'inscrire. dans la suite de notre prochaine niche qui serait dommage donc je compte sur vous pour que nous puissions dire l'essentiel le dire certes mais dans les délais donc je vous remercie infiniment de votre attention merci relativement rapidement tout en disant l'essentiel et bien cette proposition de loi nous pouvions voter sur celle-ci avant l'heure fatidique de 13h. Monsieur le rapporteur

M. le Président, Mme la Ministre, M. le Président de la Commission, mes chers collègues, nous nous sommes réunis ce matin pour examiner la proposition de loi visant à aménager la prévention des risques liés au bruit et ils sont amplifiés. Les sports mécaniques, comme vous le savez, sont de véritables patrimoine dans notre pays. Il s'agit de la troisième filière économique qui représente 2,5 milliards de chiffre d'affaires et induit 13 500 emplois. Il y a des manifestations sur 1000 circuits avec 2300 épreuves sportives pendant l'année. Donc, c'est un élément très particulier pour notre économie en général. Je vais en parler particulièrement puisque dans mon département, il y a le circuit de Longarou qui réunit de nombreux participants pendant les fêtes de Pâques chaque année. Et d'ailleurs, je salue les maires de nos garros qui sont à la tribune et qui sont venus écouter ce débat avec beaucoup d'intérêt. La proposition de loi de Nathalie Delattre, que je remercie, vise à assurer la continuité de ses activités tout en luttant contre les nuisances sonores, mais elle ne constitue pas Ils ont une entrave à la sécurité sanitaire que nous défendons tous, bien entendu. Les premiers à être conscients de cette possibilité, ce sont les fédérations sportives qui se sont engagées depuis longtemps pour réduire les nuisances sonores en améliorant la technicité sur les moteurs. De même, les fédérations des motocyclistes a agi également dans ce sens. Il ne s'agit pas aujourd'hui, comme certains l'ont dit, de court-circuiter la prévention des risques liés au bruit, mais d'adapter en définitive un dispositif législatif. Comme vous le savez, avant 2017, les circuits automobiles étaient régis par les fédérations nationales du sport automobile et des motocyclistes. Le préfet pourrait adapter dans chaque manifestation des règles spécifiques dans le cadre de ces éléments. Le décret de 2017 dit anti-bruit a été pris sans consulter les acteurs de la filière et, en définitive, mettre à l'exergue les dispositions générales relatives aux bruits de voisinage et autres que nous connaissons tous. Un circuit de vitesse, il faut le savoir, n'est pas un voisin comme les autres. Il ne faut pas laisser planer une épée de dame aux clés sur les organisateurs et sur les communes qui sont propriétaires ou concessionnaires de circuits automobiles. Il s'agit aujourd'hui de les sécuriser. C'est la raison pour laquelle il faut concilier d'une part les activités des circuits automobiles et, bien entendu, la protection de la santé humaine. La Commission qui a partagé cet avis à chercher, comme le faisons aujourd'hui, à sécuriser juridiquement le dispositif, clarifier le champ d'application des règles en la matière et, en définitive, de présenter un texte pragmatique et adapté pour trouver un équilibre entre l'exercice du sport automobile, la santé humaine et la réglementation dont il va avec. C'est la raison pour laquelle ce texte me paraît aujourd'hui tout à fait équilibré, tout à fait adapté, qui va donner un signal fort à l'économie du sport automobile et en même temps qui va faire vivrer, bien entendu, beaucoup de nos concitoyens, car nous savons qu'en France, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui créent du lien social en se rendant sur les circuits automobiles pour, justement, approuver la pratique de ces sports automobiles. Donc, je voudrais remercier, en conclusion, Nathalie Delattre, bien entendu de nouveau, d'être à l'origine de ce texte, remercier le président de la Commission, Jean-François Longiot, qui, dans sa grande bienveillance, a voulu me donner rapporteur, et également, monsieur Deluca, mon administrateur, qui a fait un travail exceptionnel dans cette affaire. Je vous remercie de m'avoir écouté quelques mots et en vous disant que Je pense que la plupart ou la majorité des collègues ici présents pourront soutenir cette disposition. Je vous remercie monsieur le rapporteur. La parole est maintenant à madame Amélie Oudéa-Castira, ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. A vous madame la ministre. Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission de l'Aménagement du territoire et du Développement durable, cher Jean-François Longeau, Monsieur le Rapporteur, cher Alain Dufour, Madame la Sénatrice, chère Nathalie Delattre, Mesdames les Sénatrices, Messieurs les Sénateurs, La France est une grande nation de sport. Et si elle l'est devenue en acclimatant un certain nombre de disciplines, notamment celle née outre-manche, à commencer par le football, le rugby, elle a également à plusieurs reprises été pionnière. C'est le cas avec le sport automobile pour lequel elle n'a jamais cessé d'être à la pointe de l'innovation, tout à la fois technologique comme en témoignent les moteurs hybrides, mais aussi sociétal, à l'image de l'introduction de la ceinture de sécurité. Et c'est ainsi que les sports mécaniques sont devenus une passion et une mythologie bien française, comme l'illustrent les 1200 circuits qui accueillent chaque année plus de 2300 épreuves automobiles et motocyclistes, mais aussi les 160 000 licenciés et les 130 000 bénévoles qui chaque semaine, partout en France et notamment dans les territoires ruraux, font vivre et rayonner ces événements. Un rayonnement qui a d'ailleurs de longue date dépassé les seules frontières de l'Hexagone, tant les noms de Manicourt, Paul Ricard et bien sûr des 24 heures du Mans se sont fait une place à part dans la grande épopée du sport mondial. Aujourd'hui, en envisageant à haute voix de retrouver un grand prix de Formule 1 chez elle, c'est cette grande histoire que la France entend poursuivre, avec la ferme volonté de continuer à concilier et à enrichir ces liens entre la passion des courses, l'innovation technologique, le développement durable et la protection de la santé publique. Voilà pourquoi, madame la sénatrice, cher Nathalie Delatt, je tenais à vous remercier d'avoir pris cette initiative parlementaire avec plusieurs de vos collègues et de manière transpartisane, dont l'objectif n'est pas, comme vous l'avez rappelé lors des travaux en commission, de placer les sports mécaniques en dehors de tout cadre en termes de prévention du bruit excessif pour les populations, mais bien d'essayer de trouver le meilleur dispositif juridique possible, c'est-à-dire un dispositif pragmatique, responsables, pleinement applicables pour permettre à ces activités de continuer à faire rayonner nos territoires dans lesquels elles sont souvent implantées de longue date tout en continuant de s'inscrire dans une dynamique de réduction de leur empreinte sur notre environnement au sens le plus complet de ce terme. Or, à l'heure actuelle, comme vos travaux l'ont démontré, le cadre juridique, celui issu du fameux décret bruit du 7 août 2017, marque une double impasse, disons-le sincèrement, dans sa philosophie comme en pratique. Dans sa philosophie d'abord, ce décret résulte en effet d'une disposition de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, mais qui a été adoptée sans concertation préalable avec les acteurs sportifs ni études d'impact. Il a donc intégré ce décret du jour au lendemain les sports mécaniques dans le champ des règles d'émergence fixées par le code de la santé publique et ce nouveau cadre législatif et réglementaire a été imposé à l'ensemble des circuits sans mesure transitoire les plaçant dans une situation particulièrement délicate alors même qu'ils étaient déjà régis par des règles techniques de la fédération des fédérations concernées mais aussi par des prescriptions relevant de leur homologation par le préfet ou le ministre de l'Intérieur. Cette erreur de méthode, hier, conduit aujourd'hui à une impossibilité pratique d'application de la réglementation par le secteur. Soumis en droit au respect de la règle d'émergence, soit la différence entre un bruit ambient, bruit durant l'activité, et un bruit résiduel, le bruit sans l'activité, les circuits sont bien souvent, malgré eux, pris au piège. Ainsi, qu'il soit en milieu urbain ou éloigné des habitations, le circuit est rarement en mesure de respecter le cadre réglementaire. En pleine ville, l'activité du circuit impacte nécessairement son voisinage immédiat, qui s'est souvent installé postérieurement à la création de l'équipement sportif. Le circuit d'Albi en est le parfait exemple, comme l'explique souvent la maire d'Albi, Stéphanie Guirauch-Aumeil. En zone rurale, le bruit résiduel étant particulièrement faible, la règle d'émergence est mécaniquement impossible à respecter. Dans cette soustraction entre le bruit ambiant et le bruit résiduel, mesurée dans les logements d'habitation du voisinage, vous voyez soit le premier terme est considéré comme trop élevé, soit le second comme trop bas, plaçant les circuits dans cette impossibilité pratique d'application de la législation. De même, certaines compétitions de premier plan, comme les 24 heures du Mans ou encore le bol d'or, ne peuvent respecter les règles d'émergence différentes entre la période durene et la période nocturne, auxquelles les compétitions sont pourtant assujetties de plein droit du fait du décrébuit. Enfin, des circuits plus modestes, jusqu'au grand prix de France de MotoGP, de nombreuses situations soulèvent les mêmes difficultés. Face à ces règles élargies au sport mécanique, nous constatons les difficultés de la filière qui se retrouvent ainsi dans un flou juridique, qui pénalise avant tout les autorités publiques, au premier rang desquels les collectivités territoriales, qu'elles soient propriétaires ou gestionnaires de certains circuits, mais aussi l'État dont la responsabilité peut être invoquée pour indemniser les exploitants ou les collectivités ayant investi dans ces circuits. Et au quotidien, face à ces difficultés, ce sont nos préfets qui se trouvent dans une position là aussi complexe en étant à la fois les autorités homologuant la plupart des circuits et celles chargées aux côtés de nos maires d'assurer la police de l'environnement. Avec pour ces règles des conséquences très concrètes puisqu'au-delà de remettre en question l'organisation de nombreuses compétitions, leur non-respect entraîne pour l'organisateur des sanctions pénales élevées. Je tiens à souligner que les deux fédérations délégataires de services publics, la fédération française de sport automobile et la fédération française de motocyclisme, n'ont pas attendu le décret bruit et la menace qu'il fait peser sur leurs disciplines pour prendre conscience de leurs responsabilités en matière de tranquillité publique et de préservation de la santé. Depuis le début des années 2000, elles travaillent en effet à une réduction du bruit généré par leurs activités, la FFSA, a d'abord adopté une politique ferme visant à réduire drastiquement le bruit à la source des véhicules avec la réduction de plus de 20 décibels sur les 20 dernières années. De son côté, la FFM a également initié un travail important depuis 2009 avec une baisse des émissions sonores qui représentera en 2024 de 5 à 7 décibels pondérés. Selon les disciplines, étant entendu qu'une réduction de 3 dBa revient à diminuer l'intensité sonore ressentie par deux. Rappelons d'ailleurs que cet engagement responsable de nos fédérations, auquel je suis particulièrement attachée, place la France à l'avant-garde mondiale, s'agissant de la mutation de la pratique des sports mécaniques. C'est en France que que la première compétition automobile électrique sur circuit s'est déroulée dès 2009 et qu'un véhicule électrique a participé pour la première fois à une compétition sur route en septembre 2020. De leur côté, plusieurs disciplines sportives ont d'ores et déjà opéré leur mutation énergétique en évoluant vers des carburants décarbonés à l'instar de la Formule 4. Plus largement, la FFSA et la FFM se sont engagés dans une démarche plus durable en se fixant un objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050 et en lançant dès 2022 le premier baromètre environnemental des sports mécaniques dont les résultats me seront très prochainement présentés. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, je considère qu'il est tout à l'honneur de l'initiative parlementaire de rechercher ce nouveau point d'équilibre qui permettrait de pérenniser un secteur automobile fleurant de notre paysage sportif. et économique nationale tout en protégeant la tranquillité publique et la santé humaine. Objectif de conciliation que je partage pleinement. Le dispositif proposé demeure probablement encore perfectible et ce sera tout l'objet de ce débat parlementaire. Au-delà de l'intitulé de la proposition de loi et du processus de consultation préalable avant adoption du décret permettant d'en assurer l'application qui font encore débat comme nous le verrons dans cette discussion. Je m'interroge aussi sur la nécessité d'exposer plus explicitement la nature des dérogations qui seraient ainsi fixées aux codes de la santé publique mais aussi de préciser la nature des prescriptions particulières auxquelles devront être encore soumis dans cette hypothèse les sports mécaniques en renvoyant le cas échéant au pouvoir d'appréciation des autorités préfectorales. Dans ce cadre, je m'engage à mener un travail spécifique pour qu'ensemble et aux côtés de nos deux fédérations délégataires, nous continuions à améliorer le dispositif que vous proposez et que nous trouvions les meilleurs équilibres en nous appuyant en tant que de besoin sur les préfets directement concernés tout en tirant parti de l'éclairage supplémentaire qui sera apporté par la remise en décembre du baromètre environnemental de la filière des sports mécaniques. Pour toutes ces raisons, s'agissant du texte aujourd'hui débattu en séance, le gouvernement s'en remettra à la sagesse du Sénat. Mesdames et messieurs les sénateurs, en nous appuyant sur votre reconnaissance inégalable de nos territoires et votre approche du droit résolument tournée vers la pratique, je suis persuadée que nous parviendrons à concilier de la manière la plus efficace et adaptée possible nos deux impératifs, pérennité des sports mécaniques, protection de la tranquillité et de la santé publique. Et vous pouvez compter sur moi pour mobiliser l'ensemble des acteurs et appeler chacun à ses responsabilités en faveur de cet objectif de progrès, appuyé sur un devoir d'exemplarité, deux horizons sur lesquels nous n'avons pas le droit de décevoir nos compatriotes. Je vous remercie. Dans la suite de la discussion générale, la parole est maintenant à Monsieur André Guiol pour le groupe du Rassemblement démocratique et démocrate Dans Merci Président. Monsieur le rapporteur, Madame la Ministre, mes chers collègues. L'entrée en vigueur du décret relatif à la prévention des risques liés au bruit a fait basculer l'ensemble des activités du sport mécanique dans le droit commun des simples bruits de voisinage. S'il était nécessaire de façon générale de mieux protéger les populations des risques liés au bruit généré par l'ensemble des activités humaines, et plus particulièrement de les épargner des nuisances sonores produites par les comportements souvent illicites et agressifs, comme ça a été souligné à travers les rodéos urbains, auxquelles les populations sont soumises. Cette proposition de loi déposée par la sénatrice Nathalie Delattre vise à aménager spécifiquement les règles qui régissent en la matière les fédérations de sports mécaniques et les gérants des circuits automobiles. En effet, sans distinction ni discernement, ces acteurs du sport mécanique se trouvent à la portée de plaintes émanant de riverains ou de collectifs associatifs et sont exposés à des poursuites pénales disproportionnées au regard des services rendus à la société. Il pourrait pourtant apparaître inoporteux de soutenir, en tout cas de favoriser, la poursuite des sports mécaniques qui reposent encore aujourd'hui sur la performance des moteurs thermiques, alors que dans le même temps, la société s'est engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est ainsi qu'elle développe une industrie décarbonée qui a le privilégi des transports électrifiés collectifs ou covoiturés et que nous assistons à la montée en puissance, ça a été dit, de courses automobiles à propulsion électrique qui contribueront à leur tour à faire à leur tour à faire progresser cette technologie en termes de performance, de sécurité et de fiabilité. Ces avancées technologiques bénéficieront bien entendu à l'ensemble du parc automobile qui pèse encore aujourd'hui lourdement dans la production du gaz à effet de serre tout en contribuant à réduire globalement les nuisances sonores qui nous préoccupent aujourd'hui, ça a été dit. En effet, rappelons que le sport mécanique dont la filière génère 13 500 emplois et pèse un impact économique de 2,5 milliards d'euros ont largement contribué jusqu'à ce jour à réduire la pollution des moteurs thermiques tout en augmentant par ailleurs de façon considérable les performances mécaniques et leur fiabilité au point qu'ils sont devenus aujourd'hui la motorisation par excellence de presque toutes les activités humaines. Citons les transports terrestres, les maritimes, le génie civil, le secteur militaire, sans oublier l'utilisation du groupe électrogène. C'est le groupe électrogène qui alimente encore de façon nombreuse les îles et les fermes isolées et qui, par leur fiabilité, vient en secours de l'alimentation électrique des hôpitaux, des centrales nucléaires et de tout le secteur industriel. C'est grâce notamment à une grande partie au progrès technologique généré par les sports mécaniques et à leur moteur thermique qu'on le doit. Les progrès générés par cette activité qu'il convient par cette PPL de préserver ont également et considérablement contribué à améliorer la sécurité routière. On peut citer l'amélioration de la tenue de route par la qualité des pneumatiques et par l'efficacité des suspensions, par la mise au point des organes de sécurité comme les ceintures de sécurité, la consolidation et l'indéformabilité des habitacles et les freinages ABS. Mes chers collègues, comme dans beaucoup de domaines, notre aventure humaine est amenée en permanence à arbitrer entre deux objectifs apparemment antinomiques. D'un côté, la nécessité de maîtriser l'évolution climatique à laquelle nous sommes confrontés et de faire preuve, par ailleurs, de courage durant cette transition afin de poursuivre nos utiles activités économiques parfaitement encadrées. C'est une des vertus de cette PPL. pour traduire cette situation, je rappellerai la phrase éclairante de Jean Jaurès, qui a déjà été citée ce matin. Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. soucieux de nourrir cette vertu. La majorité de mes collègues du RDSE approuveront cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci Monsieur le Sénateur. Décidément, Jean Jaurès est à l'honneur. Maintenant, Madame Nadejavé pour le groupe RDPI du Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants va s'exprimer et ce pendant cinq minutes. La sénatrice. Bonjour Monsieur le Président. Madame la ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, cher Nathalie Delattre, Mes chers collègues, La proposition de loi de notre collègue Nathalie Delattre entend aménager la prévention des risques liés au bruit et au son amplifiés en soumettant les sports mécaniques à des prescriptions dérogatoires. Celles-ci devront concilier leurs pratiques avec la protection de la tranquillité du voisinage et de la santé humaine. Les modalités d'application seront à préciser dans un décret du Conseil d'État. Pour faire suite à la loi de modernisation du système de santé voté en 2016, le décret du 7 août 2017 est venu définir en ce domaine l'ensemble des mesures obligatoires dans les lieux ouverts au public ou recevant du public ainsi que celles des riverains. plus spécifiquement concernant les activités des sports mécaniques. Cette mesure est venue modifier le niveau sonore applicable en soumettant les circuits aux droits communs des bruits de voisinage. Depuis lors, les circuits de sports mécaniques sont désormais soumis à deux réglementations complémentaires. d'une part les règles techniques et de sécurité édictées par les fédérations délégataires qui fixent le niveau sonore à la source et d'autre part les articles précités qui fixent les émergences sonores émises par l'activité des circuits lorsqu'elles atteignent les habitations riveraines. Un arrêté en 2023 est venu à son tour apporter des précisions. Dans ce cadre, nouvellement défini, le constat est dressé dans la proposition de loi que les circuits de sport mécanique se trouvent désormais soumis à des règles disproportionnées, voire parfois inapplicables. Plusieurs lieux en France se retrouvent ainsi dans l'incapacité de respecter la réglementation en vigueur, y compris le circuit de Nevers-Manicour ou encore le circuit des 24 heures du Mans qui doit s'adapter à deux niveaux de réglementation, celui entre la période d'urne et la période nocturne. Cette situation apparaît en effet difficilement conciliable avec les activités concernées. le risque évident de contentieux préoccupe les fédérations sportives délégataires en raison de l'insécurité juridique et technique dans laquelle elles se trouvent désormais. Pour répondre à cette problématique, le texte propose donc de soumettre les sports mécaniques à des prescriptions particulières. Nous rappelons ici qu'il y a un apératif à lutter contre la pollution sonore et la Commission européenne l'a encore récemment rappelé. Mon groupe, s'il votera majoritairement en faveur du dispositif proposé, souhaite que les efforts des constructeurs et des organisateurs se poursuivent évidemment. et que le décret prévu par le texte fixe une trajectoire certes practicable mais ambitieuse en matière de gestion des bruits. J'ai d'ailleurs pu prendre connaissance de certaines avancées en la matière, notamment dans le domaine du motocyclisme, qui ont accompli d'importants progrès pour réduire les nuisances sonores. Je veux également profiter de cette discussion générale pour saluer l'engagement des professionnels du spectacle vivant qui font face eux aussi à d'importantes contraintes en la matière et à une réglementation sonore ambitieuse. Autour de 3 000 festivals musicaux sont impactés en France. Alors que les professionnels concernés doivent relever un grand nombre de défis techniques, les expérimentations sont menées afin de concilier la qualité de l'expérience sonore et le respect de l'environnement. Ces démarches complexes mais volontaristes préfigurent les festivals de demain. Je vous remercie. Merci Madame la Sénatrice. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Madame Nicole Bonnefoy pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le texte qui nous est présenté ce matin par notre collègue Nathalie Delattre vise à déroger aux droits communs en matière de prévention des risques liés au bruit émis par des circuits automobiles. Pour rappel, ce décret a été pris dans la continuité de l'article 56 de la loi de Marisol Touraine sur la modernisation de notre système de santé qui permettait de renforcer la protection des riverains exposés au bruit. L'impact des nuisances sonores sur la santé et son coût social est clairement démontré par une récente étude de l'ADEME. Les nuisances sonores sont à prendre en compte en termes de santé environnementale et de santé humaine. De manière identique, nous avions été alertés par la difficile application du décréton pour les festivals. Je note également les efforts des fédérations sportives pour s'adapter en organisant des compétitions de véhicules électriques ou encore un baromètre environnemental des sports mécaniques. Il est impérieux d'aller plus en avant dans cette voie car ces activités de loisirs automobiles ont de forts impacts en matière de consommation d'énergie fossile. Sans méconnaître bien sûr l'importance de ce secteur, il est cependant nécessaire d'encadrer le dispositif qui nous est proposé afin que les rêverains se sentent suffisamment protégés de toute dérive sonore ouverte par un nouveau décret. Un outre, si nous pouvons entendre les objectifs des auteurs de la proposition de loi, Il ne faudrait pas que notre assemblée s'empêche de veiller à ce que des garde-fous soient clairement posés. A ce titre, nous avons déposé trois amendements qui garantissent, selon nous, un meilleur encadrement du dispositif. D'abord, la consultation du Conseil national du bruit à la rédaction du décret. En effet, la consultation de cette instance dans l'élaboration du décret nous paraît indispensable pour la bonne raison qu'il est composé de représentants des collectivités locales, des organisations syndicales, des personnalités qualifiées et des représentants des différents groupements, associations et professions concernés par les problèmes de lutte contre le bruit et d'amélioration de l'environnement sonore. Certes, le Conseil national du bruit détient un pouvoir d'auto-saisine, mais les choses vont mieux en le disant, mes chers collègues, surtout dans le cadre de ce texte qui laisse peu de marche de manœuvre parlementaire que nous sommes, puisque le texte renvoie au pouvoir réglementaire le soin de réviser le décret. En second lieu, poursuivant l'objectif de sécuriser le dispositif, nous défendons l'introduction d'un nouvel article qui permettra d'évaluer au moyen d'un rapport remis au Parlement la dérogation permise par cette proposition de loi. Il me semble très important que nous puissions assurer le suivi de décisions que nous prenons ici, car le sujet ne concerne pas uniquement la filière des sports mécaniques, mais aussi les riverains. Un rapport d'évaluation permettra de veiller à la bonne application et à un équilibre entre les besoins de l'ensemble des parties prenantes. Enfin, nous vous proposerons de modifier l'intitulé de la proposition de loi dans le but de clarifier l'objectif de ce texte. L'ensemble de nos propositions d'amendement vise donc à trouver un meilleur équilibre entre la préservation de la filière des sports mécaniques et la préservation de la santé humaine et la protection du voisinage. J'avoue ne pas comprendre les positions rigides exprimées par le rapporteur en commission vis-à-vis de ces amendements. Vous avez dit tout à l'heure monsieur le rapporteur avoir cherché à concilier tous les avis, ce n'a pas vraiment été le cas jusqu'à maintenant. J'espère que la discussion qui s'ouvre permettra d'améliorer ce texte qui à ce stade ne demande aucune contrepartie aux bénéficiaires de la dérogation prévue. Par ailleurs, à la suite d'une question écrite de l'un de nos collègues, le ministère avait indiqué qu'un groupe de travail avait été mis sur pied et une réunion interministérielle s'est tenue en octobre 2021 en présence de la fédération française de motocyclistes et de la fédération française du sport automobile. Pourriez-vous nous dire, Madame la Ministre, nous en dire plus sur les avancées de ce groupe de travail ? Avez-vous d'ores et déjà prévu des aménagements du décret et dans quel sens ou en sont les conclusions ? Ces éléments auraient peut-être été très utiles pour éclairer notre débat et rendraient peut-être de fait ce texte assez inutile au regard des évolutions réglementaires envisagées par le gouvernement. Pour en terminer, concernant notre position, vous l'aurez compris mes chers collègues, elle demeure circonspecte face au manque de souplesse du rapporteur, plus particulièrement en commission. Si nos amendements devaient être rejetés en séance, nous n'aurons d'autre choix que de nous opposer à la proposition de loi telle qu'elle est présentée. Merci Madame la Sénatrice. La parole est maintenant à Madame Martha de Citrac pour les Républicains et ceux pour six minutes.

Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, en tant qu'ancien membre du Conseil national du bruit, je ne peux que me réjouir de l'examen de cette proposition de loi qui nous donne l'occasion de nous exprimer sur un sujet tellement sensible pour la majorité de nos concitoyens, le bruit. Et d'emblée, je partage avec vous ma conviction que mieux différencier, mieux encadrer les risques liés au bruit est une bonne initiative. Ce n'est certainement pas créer un droit à la pollution sonore. La filière des sports mécaniques en France concerne des technologies au service d'une recherche industrielle de pointe qui s'intéresse au développement de la sécurité automobile et bien sûr au développement économique. Elle représentait il y a cinq ans encore environ 13 000 emplois et 2,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Biocarburant, hybridation, motorisation électrique, remplacement du carbone par le chanvre, télémétrie, aérodynamique, toutes ces technologies viennent initialement de la course automobile et sont maintenant érigées comme d'incontournables standards pour réussir la transition écologique. Pour saisir l'opportunité de ces innovations, il est essentiel qu'à tous les niveaux et dans toutes les disciplines, les sports mécaniques tiennent compte des évolutions de notre société et conservent un écosystème d'infrastructure dynamique. A ce titre, je salue l'emblématique circuit Jean-Pierre Beltoise de mon département, acteur engagé dans le domaine de la sécurité routière. Cependant, cette dynamique est aujourd'hui fragilisée, raison pour laquelle nous sommes réunis. En effet, les sports mécaniques pâtissent depuis 2017 de l'application d'un régime général sur la sanction des nuisances sonores. Même si l'intention de ce régime général est parfaitement compréhensible, prenons garde de ne pas menacer l'existence même d'une activité qui s'avère dynamique dans les territoires. Cette règle pourrait à terme s'avérer néfaste pour toute une filière et obéirer la France des opportunités pour son rayonnement sportif et industriel. En appliquant le droit existant, même les très vertueuses formules électriques, pourtant érigées en modèle de la compétition automobile durable, seraient en infraction. En effet, une monoplace électrique produisant environ 85 décibels, c'est un seuil suffisant de bruit d'activité pour contrevenir à la loi. Il s'agit d'un exemple parmi tant d'autres des incohérences qui parfois se glissent dans notre droit et qui pénalise ce qui est devenu un véritable laboratoire pour une industrie automobile durable et responsable. Au-delà de l'urgence climatique, les objectifs européens vers lesquels cette industrie doit tendre en matière de transition écologique et de mobilité durable nous rappellent que le temps presse. En renvoyant les sports mécaniques à un régime différencié du droit commun, nous ferions donc œuvre utile et de bon sens. Il n'est nullement question d'autoriser sans contrôle une pollution sonore active, mais de mieux encadrer les pratiques. particulièrement sensible à la problématique du bruit, je souhaite qu'un chemin de crête équilibré soit trouvé. Nos concitoyens et riverains des circuits ont, comme chaque Français, droit à la tranquillité publique. Le sport mécanique n'est pas le seul domaine où la lutte contre la pollution sonore peut se concilier avec des objectifs économiques et écologiques. Bien qu'étant en dehors du champ de la loi de 2016, le transport aérien connaît lui aussi des adaptations aux réalités locales en cas de survol à basse altitude des zones habitées. C'est un problème que les Yvelines connaissent bien et j'ai d'ailleurs plusieurs fois interrogé le gouvernement sur la mise en œuvre des trajectoires d'approches aériennes dites en descente douce. Cette alternative semble convenir à tous les acteurs, preuve que s'adapter à certaines réalités sectorielles est souvent une solution de bon sens. Malgré tout, le bruit est devenu un démo du monde moderne. L'intensification du transport routier, aérien, ferroviaire, le bruit des activités économiques, la généralisation des casques et écouteurs audio, tout cela fait peser sur notre système auditif de fortes contraintes. Avec la pollution lumineuse qui est souvent associée au bruit, ce n'est pas sans conséquence sur notre santé, sur la biodiversité ou sur les milieux naturels. Rendons-nous compte, l'audition est une des fonctions de l'organisme qui ne cesse jamais. Le bruit entraîne pour l'homme des troubles du sommeil, engendre des pathologies cardiovasculaires sérieuses et des dommages auditifs parfois irréversibles. Ces problématiques doivent être considérées avec le plus grand sérieux. Plus généralement, je salue le travail de tous les acteurs qui se mobilisent dans le domaine de la lutte et de la prévention contre les nuisances sonores. Je sais les élus locaux et les services de l'Etat particulièrement engagés, notamment à travers les plans d'exposition au bruit. Mais le problème n'est pas que politique ou administratif. Il y a un travail de sensibilisation important à réaliser auprès de nos concitoyens, de même que certains secteurs comme celui de la construction devront prendre leur part. On entend beaucoup parler de l'isolation thermique des bâtiments, mais peu de l'isolation sonore. Comme la performance thermique, la résilience acoustique d'âme bien fait partie du diagnostic immobilier. On l'oublie trop souvent. Mes chers collègues, ce texte améliorera la prévention et la lutte contre les nuisances sonores issues des sports mécaniques. Comme souligné à plusieurs reprises, il ne vise nullement à créer une exception juridique, mais bien à adapter un dispositif trop large qui ignore la réalité des contraintes sonores liées aux sports mécaniques. Le droit à la différenciation ne rime nullement avec l'octroi de privilège. Toutes ces raisons, vous l'avez deviné, nous voterons cette proposition de loi. Il restera évidemment à être vigilant sur son application réglementaire car le double enjeu économique et sanitaire de ce texte devra être respecté. Je vous remercie. Merci madame la sénatrice. La parole est maintenant à monsieur Cédric Chevalier pour le groupe Les Indépendants. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, sur l'ensemble de nos territoires, les courses automobiles sont de réels lieux d'échanges et de rencontres. Bien sûr, la Formule 1 ou encore les 24 heures du Mans sont les vitrines de ces sports mécaniques, mais nous avons tous dans nos départements un rallye ou des compétitions auto et moto sur les nombreux circuits automobiles que compte la France. C'est une partie intégrante de notre culture. Sans vouloir paraître chauvin, je vous citerai pour ma part le célèbre circuit de gueux proche de Reims et classé au patrimoine monumental français ou le rallye des Vins et de Champagne qui a vu débuter Sébastien Loeb dans cette catégorie ou enfin le passage certaines années dans notre beau département du rallye Monte Carlo historique. A titre personnel, si vous le permettez, j'ai été bercé par les exploits de mon arrière-grand-père Charles Delphos, constructeur et pilote automobile dans les années 20 qui a notamment affronté les 6 heures des roues de pavé avec des voitures dont il avait conçu Les châssis. Aujourd'hui, et comme l'ont déjà évoqué les orateurs précédents, les sports mécaniques sur circuit sont soumis à des strictes restrictions en matière sonore qui ne correspondent pas à la réalité de ces pratiques, alors même que depuis de nombreuses années, les fédérations sportives automobiles œuvrent à la réduction de toute forme de pollution, y compris sonore. Les progrès sont sous nos yeux et cette PPL l'explique très bien. J'en profite pour saluer le travail du rapporteur et de l'auteur et de notre commission sur ce texte. Nous avons en effet été très attentifs au développement et aux orientations que nous souhaitions impulser pour le secteur automobile. De manière générale, nous avons voulu instaurer un cadre permettant à la fois de réduire les nuisances que provoquent les véhicules routiers tout en laissant aux inventeurs la possibilité d'innover en la matière. Parce qu'il est essentiel de desserrer l'étau quand il est trop pressurisant ou qu'il l'est inutilement, nous avons eu à mettre en place des dispositions pragmatiques pour les sports automobiles. Comme cela a été rapporté, il n'est pas question de mettre en place un droit à la pollution sonore, mais bien de trouver une voie équilibrée en permettant le développement et la pratique de ce sport tout en tenant compte des contraintes extérieures et d'une usance possible. Toutefois, permettez-moi, il est à noter que les circuits automobiles ne sont pas sortis de terre ces dernières années et la plupart d'entre eux existent en effet depuis un certain temps. Que les riverains se plaignent maintenant des niveaux sonores peut paraître surprenant. Nous ne sommes pas dans un film d'Yves Robert où des quadrats achètent une maison de campagne au bord d'un aéroport un jour de grève des avions. Plus sérieusement, ce texte soulève une question plus profonde. Alors que nous sommes en pleine transition et particulièrement en pleine réflexion sur nos modes de transport, il faut rappeler que les avancées techniques développées dans le sport auto se répercutent sur l'ensemble de l'industrie automobile et servent à tous les conducteurs. Je ne reviendrai pas sur les chiffres économiques de la filière, ni même les milliers d'emplois créés pérennes. J'aimerais simplement évoquer l'excellence de la France dans ce domaine, car nous sommes reconnus à travers le monde pour notre savoir-faire en la matière. Je vous rappelle que le moteur turbo a été développé grâce à la Formule 1. Le système anti-blocage des roues, plus connu sous le BS aussi, il sauve bien les vies depuis qu'il est sur nos voitures de série. Le système de récupération d'énergie cinétique vient également tout droit des circuits de Formule 1. Quant aux freins de disque, ils ont été d'abord présentés lors des 24 heures du man. En bref, ce qui se passe sur nos circuits de sport mécanique est un véritable accélérateur d'innovation et le travail sur les nuisances sonores en fait partie. Il faut donc trouver une position équilibrée entre la pratique de ces sports mécaniques et les nuisances sonores qu'ils engendrent. Je rappelle que les filtres intelligents placés au niveau des moteurs réduisent les bruits. De nombreuses améliorations ont été effectuées de ce côté. Pour toutes ces raisons, le groupe Les Indépendants, investi par le Progrès et l'Innovation, trouve ce texte équilibré et votera donc en sa faveur. Je vous remercie. Merci, monsieur le Sénateur. La parole est maintenant à madame Nadia Sologoub pour le groupe Union Centriste et ce pour 6 minutes. Madame la Sénatrice. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues, dans cet univers plein de bruit et de fureur, c'est le bruit des uns qui provoque la fureur des autres, nous dit Antoine Blondin. Difficile de trouver citation plus appropriée pour introduire le texte qui nous occupe aujourd'hui. Pour autant, bruit et fureur sont relatifs à des lieux et des circonstances. Un bruit insupportable ici peut être jugé tout à fait acceptable là-bas. C'est cette réalité à géométrie variable qui est aujourd'hui interrogée. Dans un souci de protection de la santé publique, le législateur a souhaité, par un décret pris le 7 août 2017, établir une règle de protection des riverains, des risques liés, je cite, au bruit et au son amplifié. Le texte définit des niveaux sonores à respecter par des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés. Il détermine également des mesures de protection individuelle des risques auditifs tels que l'information du public, la mise à disposition de protection auditive et la mise en place de dispositions permettant le repos auditif. Les seuils sont fixés en décibels dits pondérés, des niveaux de pression acoustique maximum sur une durée déterminée. Ces dispositions concernent des activités impliquant la diffusion de sons à des niveaux sonores élevés tels les festivals. Le décret comporte également un volet concernant les lieux hébergeant des activités susceptibles d'occasionner la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés en prenant cette fois en compte un critère d'émergence, vous nous l'avez dit Madame la Ministre, de bruit, c'est-à-dire la différence entre le niveau de bruit ambiant comportant le bruit particulier mis en cause et le niveau de bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels. Curieusement, on trouve dans ce décret des dérogations pour les bruits provenant des infrastructures de transport et des véhicules qui circulent, des installations particulières de la défense nationale, des installations nucléaires de base, des installations de transport et de distribution d'énergie, des mines, des carrières et de certains ICPE. De même, pour une raison qui m'est inconnue, des lieux hébergeant des activités bruyantes situées à Saint-Barthélemy. Ce cadre, qui se voulait de bon sens, trouve des limites logiques et il faut évidemment des dérogations. Mais cela induit des incohérences. Ainsi, dans le cadre dérogatoire, le bruit émis par un véhicule sur une infrastructure routière n'est pas plafonné. comme si on considérait qu'il ne représente pas de risque pour la santé des riverains. Depuis l'apparition du décret bruit de 2017, le même bruit émis par le même véhicule peut être interdit si les produits dans l'enceinte d'un circuit automobile est ceci pour protéger la santé de ces riverains. Comme si la santé des riverains d'une autoroute comptait moins que la santé des riverains d'un circuit automobile. Ce n'est pas anecdotique car, au-delà d'être incohérent, ce système a de graves conséquences pour le sport automobile. Il représente une menace certaine pour les manifestations et, par suite, les circuits qui se trouvent désormais dans une situation juridique fragile. Nous sommes plusieurs sur ces bancs à mesurer le rayonnement des circuits automobiles, leur effet d'entraînement sur les entreprises locales qui se constituent souvent en pôles techniques, économiques et de formation, véritables creusets de recherche pour nos territoires. Nous constatons également, pour le pratiquer au quotidien, qu'un fonctionnement dynamique régulier engendre une attraction touristique et ruisselle sur tous les lieux d'hébergement touristique. Je vous en parle savamment car, élu de la Nièvre, département rural peu connu, combien de fois ai-je constaté que l'unique moyen de faire identifier mon territoire, c'est de citer le circuit de Nevers-Manicourt et le vin de Pouilly, je dois bien vous l'avouer. Ainsi, certaines populations sont venues s'installer chez nous en raison des occasions professionnelles générées par le circuit. Personne n'a acheté une maison sans remarquer sa présence à proximité. Tous les riverains le sont en connaissance de cause. Le maire me confirme que le circuit tout proche est pour sa commune un atout inestimable et non pas une source de conflit ou de tension. Il a fait venir plus d'habitants qu'il en a fait partir. Il me livre même deux anecdotes révélatrices. Habitué qu'il ait à entendre des moteurs, il me dit reconnaître à l'oreille lorsque c'est une F1 des années 70 qui tourne tant elle est plus bruyante qu'une voiture contemporaine. Ce qui en dit long sur les progrès réalisés dans le domaine par le sport automobile en général. Il me dit aussi qu'on a installé sur sa mairie un ma de mesure de bruit qui lui a surtout permis de constater que les nuisances proviennent surtout des fortes circulations sur l'autoroute tout proche. Madame la Ministre, mes chers collègues, en tout état de cause, il faut de la mesure. Alors, citation pour citation, comme nous le dit Sénèque, ayons le souci de séparer les choses du bruit qu'elles font. C'est ce que nous faisons en autorisant la circulation sur les actes routiers et le fonctionnement d'équipements industriels pourtant bruyants. Considérant l'apport indéniable du sport automobile, ses retombées économiques, les avancées technologiques qu'il nous offre, permettons à nos préfets de reprendre la main et de pouvoir localement avec discernement autoriser ce qui peut l'être. Permettons aux acteurs locaux, élus et dirigeants d'équipements sportifs de mettre en place une solution qui vaut mieux que tous les décrets, la discussion, l'écoute et le travail en bonne intelligence. Merci donc à notre collègue Nathalie Delattre d'avoir porté ce texte et à mon collègue Alain Dufour du groupe Union Centriste de l'avoir si bien rapporté. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, le groupe Union Centriste votera pour cette proposition de loi le pied au plancher. Merci, merci beaucoup madame la sénatrice. La parole est maintenant à monsieur Jacques Fernic pour le groupe écologiste solidarité et territoire pour quatre minutes. Merci, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. La pollution sonore, c'est sans doute une des pollutions les plus négligées. Pourtant, ces impacts sanitaires sont bien démontrés. L'OMS nous le dit, le bruit c'est le second facteur environnemental provoquant le plus de dommages sanitaires juste après la pollution atmosphérique. C'est de l'ordre de 20% de la population européenne, ce qui fait quand même près de 100 millions de personnes, qui se trouve exposée de manière chronique à des niveaux de bruit préjudiciables pour la santé. Ça n'affecte pas que la santé humaine, presque toutes les branches du vivant, la biodiversité, les espèces animales subissent des perturbations comportementales de reproduction, de communication en raison du bruit intense et dans un contexte global déjà délétère pour la faune, il y a donc urgence à faire moins de bruit. Il y a une étude conjointe du Conseil national du bruit et de l'ADEME qui estime le coût social total du bruit en France à 147 milliards d'euros chaque année. J'ai bien dit 147 milliards d'euros chaque année. La présente proposition de loi qui vise à accorder aux sports mécaniques sur circuit une dérogation à la réglementation anti-bruit va donc à l'encontre à contre-courant des préoccupations environnementales, des préconisations issues des rapports scientifiques, du droit européen, de nos codes de l'environnement et de la santé publique. Aujourd'hui, notre code de la santé publique protège les personnes exposées au bruit des circuits. Cette proposition de loi serait, quoi qu'on en dise, un recul de leur droit à la santé. Le groupe écologiste s'y opposera donc. Il est essentiel de maintenir, de tenir des normes sérieuses Elle s'impose au regard des problèmes de santé que provoque l'exposition à des niveaux élevés de bruit. On l'a dit, hypertension, maladies cardiovasculaires, mortalité prématurée. Ça affecte significativement la santé physique mentale, en particulier des riverains vivant à proximité des circuits de vitesse qui vont alors bien être impactés. Dans ma région, en Alsace, à Biltzheim, face au vacarme des bruits des moteurs d'accélération, de freinage, du circuit de l'anneau du Rhin et aussi face aux effets collatéraux des voitures et motos qui traversent sans retenue les villages voisins du circuit, ça va jusqu'à Pfaffenheim, nombre de riverains sont contraints d'une certaine façon de cocher régulièrement le calendrier des événements du circuit pour se débrouiller, pour quitter à chaque fois leur domicile. ou est dans de telles conditions, monsieur le rapporteur, la création du lien social. Donc il paraît intolérable de pas protéger nos concitoyens grâce à des normes sérieuses. Le décret anti-bruit 2017, ce sont des normes sérieuses. Bien sûr, bien sûr les circuits provoquent de la ferveur populaire, de la passion, de l'engouement. Certes, on reconnaît l'importance économique, sociale, culturelle des sports mécaniques pour les territoires concernés. Ils ne doivent pas être pour autant pratiqués au détriment de la santé publique et de la protection de l'environnement. Quant à l'argument que j'ai entendu... de l'antériorité de ces circuits vis-à-vis de riverains qui se seraient localisés en connaissance de cause, donc postérieurement. Je crois que cet argument, il relève d'une logique à laquelle nous, les écologistes, on a l'habitude de se confronter depuis des décennies. Il témoigne, et si on y réfléchit bien, d'une singulière conception des principes républicains et de la valeur accordée aux codes de la santé publique et de l'environnement. Quand un ancien pilote Directeur des Curies, ancien responsable de circuit, déclare sans embâche tout récemment que, je cite, « La moitié de l'intérêt de ce sport vient du bruit du moteur. Il nous fait crûment comprendre combien ces sports motorisés doivent se transformer à l'heure où les engins thermiques sont engagés dans une transition inéluctable vers l'électrique, combien la culture qu'ils entretiennent doit se remettre en question, évoluer. Les sports mécaniques ont aussi leur transition à mener. Certains en ont d'ailleurs tout à fait conscience. Si nous votons cette proposition de loi, je crois que nous ne les y aiderons pas. Nous n'y contribuerons pas. monsieur le sénateur. La parole est maintenant à madame Marie-Claude Varayas pour le groupe communiste républicain citoyen écologiste Canachy. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. La prévention des risques liés au bruit est un enjeu important, notamment en matière de santé publique. Le bruit peut causer des troubles du sommeil, des maladies cardiovasculaires, des pertes d'audition, mais aussi tout simplement dégrader la qualité de vie de nos concitoyens. Un rapport de l'ONU publié en 2022 estime que l'exposition durable au bruit ambiant contribue à 48 000 nouveaux cas de cardiopathie et provoque 12 000 décès prématurés par an en Europe. 22 millions de personnes en Europe souffrent de nuisances sonores chroniques. Ces chiffres illustrent bien cette occupation importante qui a poussé certaines communes à expérimenter les radars anti-bruits. Si la plupart des réponses apportées s'intéressent à la source du bruit, ce sont aussi les politiques d'aménagement, notamment favorisant la présence d'arbres en ville, de parcs par exemple, ou encore l'isolation des bâtiments qui permettent d'intervenir plus efficacement contre la pollution sonore. Nous devons aller ensemble dans ce sens, vers un apaisement des ambiances, en ville comme à la campagne. L'amélioration de la qualité de vie de tous nos concitoyens est une boussole qui doit guider notre action. Aménager la prévention des risques liés au bruit, d'après l'intitulé de la proposition de loi, s'avère finalement être une réduction de la prévention de ces risques faite plus précisément au détriment des riverains des circuits automobiles. Nous comprenons bien l'enjeu de permettre aux sports automobiles et motocyclistes de vivre. Ils contribuent à l'attractivité de nombreuses communes et à leur économie. Nous n'en doutons pas. La technologie mécanique, l'enjeu des courses et l'agilité des pilotes en font un spectacle pour beaucoup de Françaises et de Français, y compris pour certains riverains de ces circuits. Toutefois, nous pensons que si des règles régissent les courses en termes de poids des véhicules, de taille, de carburant, rien n'empêche que des règles régissent aussi des normes en matière de bruit. Ces règles-là peuvent tout à fait faire partie du jeu et être prises en compte par les fédérations. Elles seront même une opportunité pour que les différents fabricants de véhicules, afin que les écuries de courses automobiles et motocyclistes apportent des innovations sur les moteurs et ainsi les rendent plus silencieux tout en étant plus performants. Ces courses sont un loisir, souvent une passion, et les passions de quelques jeunes ne doivent pas constituer une nuisance pour toutes et tous. La proposition de loi que nous examinons ce matin souhaite modifier la loi pour qu'un décret du Conseil d'État permette à ces courses d'avoir lieu au-delà des normes fixées par le décret bruit. Nous présenterons tout à l'heure un amendement afin que ce décret tienne compte de l'avis du Conseil national du bruit dont le rôle est justement de sensibiliser à ces enjeux qui semblent malheureusement ignorés par les auteurs de la proposition de loi. Donc, si cet amendement devait ne pas être retenu, comme ce fut le cas en Commission, pour le nôtre comme pour les autres, notre groupe qui souhaite préserver la santé et la qualité de vie des riverains des circuits qui tolèrent déjà des mises en sonore importantes en l'état actuel du droit, serait amené à voter contre cette proposition de loi. Je vous remercie. Nous allons examiner l'article unique et nous sommes saisis d'un amendement numéro 5 qui va être présenté par M. Fernick, sans doute. Allez-y, cher collègue. Oui, je viens de le faire par ma déclaration générale. Donc on est tenu par les délais de terminat 13 heures, donc il faut aller vite, sans faire trop de bruit quand même. Donc considérez que j'ai défendu cet amendement. Oui, Monsieur le Président, Oui, Monsieur le Président, sur cet amendement, c'est un avis défavorable, car je crois que le texte a été élaboré dans des conditions équilibrées pour permettre l'exercice des sports mécaniques et en même temps de protéger la santé la santé des hommes et la santé également de toutes les espèces. Merci. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Ministre. Président, je vous remercie. Comme je l'ai indiqué lors de la discussion générale, je crois que nous avons besoin d'avoir un débat parlementaire sur ce sujet. Aujourd'hui, on le voit, le dispositif actuel pose toute une série de difficultés pour les sports mécaniques et les circuits. Il nous faut absolument arriver à mieux concilier la pérennité pour ces sports mécaniques et les impératifs qui sont liés à la tranquillité publique, à la préservation de la santé. A cet égard, je pense que la proposition de loi, elle apporte de premiers éléments de réponse, mais elle peut encore être améliorée. Nos réflexions doivent se poursuivre. Le but, c'est d'éviter qu'il y ait des effets de bord, de ne pas remettre en cause tout un édifice construit depuis 2016, mais de trouver une réponse qui soit bien adaptée, bien proportionnée pour la question des circuits automobiles, sans détricoter, encore une fois, les choses. Au global, je m'en remets à la sagesse du Sénat concernant cet amendement tout en souhaitant sur la forme que le débat puisse avoir lieu, que les réflexions puissent se poursuivre afin de trouver les bons équilibres. Oui, merci.

de mon collègue et effectivement son efficacité pour que nous puissions rentrer dans les temps. Merci beaucoup. J'apprécie beaucoup. Merci. Mais comme vous le savez, la courtoisie est toujours de règle au Sénat. Monsieur Fernic. Une petite exception, juste pour faire remarquer que le décret date de 2017, on est fin 2023. J'entends la volonté de trouver un équilibre, que ça serait inapplicable, disproportionné, mais est-ce qu'il y a vraiment une volonté d'avancer dans ce sens-là ? Tout à l'heure, ma collègue Nicole Bonnefoy évoquait la question, je crois que c'était Patrice Jolie, auquel le gouvernement avait répondu en 2021 en disant qu'un groupe de travail était en place pour avancer sur ces questions. On n'a pas eu de réponse là-dessus. Qu'est-ce que c'est devenu ? Je remercie. Je vais mettre au voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de la Commission et un avis de sagesse de la part du gouvernement. Qui est pour cet amendement ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il n'est pas adopté. Ensuite, plusieurs amendements sont l'objet d'une discussion commune. Merci monsieur d'une discussion commune. Merci monsieur le Président, merci Madame le Ministre. Juste pour faire très rapidement, je vais faire comme le collègue Jacques Fernic, on va essayer d'être efficace et tout en restant un peu dans le timing. Bon, il nous paraît quand même assez délicat de légiférer au cas par cas, c'est vrai qu'à chaque fois qu'un problème se pose, on va apposer une loi et à partir de là, je pense qu'on n'est pas On n'est pas sorti des sollicitations des uns des autres sur l'ensemble de ce qu'on doit légiférer. Mais ce que nous proposons dans cet amendement, c'est que d'abord, il y ait un avis rendu du Conseil national du bruit, de toute façon, sur ces sujets-là, parce que je pense que le travail législatif est important, mais à un moment donné, il y a des structures qui sont absolument compétentes sur ces sujets, qu'il faut certainement d'abord consulter et avec qui il faut travailler. on ne peut pas s'en sortir malheureusement autrement et cette proposition d'ailleurs a été saluée par l'association Antibruit de voisinage qui défend quand même le voisinage des effets collatéraux des sports mécaniques et concernant le bruit c'est un sujet extrêmement sensible c'est un sujet qui est très technique et on parle d'isolation du bruit on parle de correction acoustique c'est des logarithmes à chaque fois qu'on passe 3db on double la pression acoustique et les stratégies qui sont menées pour pouvoir remédier à la pollution qu'est le bruit sont souvent très coûteuses et très contraignantes donc j'entends que les sports mécaniques qui font avancer la technologie et permettent avec des moteurs certainement moins bruyants de réduire le bruit à la source, malgré tout ce qu'il faudra mettre en place pour assurer une bonne correction acoustique et une isolation des bruits émergents sur ces sujets-là, je pense que les constructeurs et les sociétés qui gèrent les pistes vont certainement avoir beaucoup de problèmes pour les gérer sur le fond. Merci. Merci. Amendement numéro 2. Présentée par Mme Bonnefoy, je vous en prie. au sujet que nous sommes en train d'évoquer et qui peut par conséquent être parfaitement consulté. Vous allez me dire qu'elle peut s'auto-saisir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est mieux si c'est inscrit dans cette proposition de loi, rappeler la composition du Conseil national du bruit et composée de collectivités collectivités locales, des organisations syndicales, des personnalités qualifiées, des représentants des différents groupements des associations et professions concernées par les problèmes de lutte contre le bruit et d'amélioration de l'environnement sonore. Donc encore une fois, nombre de personnes qui ont parfaitement compétence pour évoquer ces sujets. Donc je ne comprends pas qu'on puisse pas inscrire dans la loi la consultation obligatoire du Conseil national du bruit. Amendement numéro 7, toujours en discussion commune, madame Ave. Il est défendu. Avis de la Commission sur ces différents amendements qui sont identiques. Oui, Monsieur le Président, c'est un avis défavorable, car on sait que le ministère de l'Environnement peut saisir le Conseil national du Brie, étant précisé aussi que le Conseil national du Brie peut saisir par lui-même. Voilà. Donc c'est un avis défavorable. Merci. Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président, un avis de sagesse sur ces différents amendements allottis pour simplement faire valoir que le texte aujourd'hui prévoit déjà la consultation pour avis de la commission nationale d'évaluation des circuits de vitesse. Cette commission, elle est aujourd'hui déjà consultée lors de l'instruction de la délivrance de l'homologation des circuits. Elle a une vraie expertise en la matière. Le Code du sport prévoit lui-même que cette commission a pour mission de vérifier que les circuits respectent les règles techniques de sécurité et aussi de proposer les dispositions qu'elle estime justifiées par les nécessités à la fois de la sécurité, de la tranquillité publique et avec évidemment la prise en compte de la lutte contre les nuisances sonores. Pour ces raisons, il me semble que l'objectif est pleinement atteint, l'objectif qui est poursuivi, il est pleinement atteint, sans qu'il y ait besoin de rajouter cette consultation obligatoire d'une autre instance. Mais je ne veux en aucun cas remettre en cause bien sûr la légitimité du Conseil national du bruit. Simplement, point de vigilance sur le fait de ne pas non plus alourdir cette procédure. Merci beaucoup. Si j'ai bien compris, votre avis est... Sagesse. Non, parce que tout a mené à penser au bout de votre explication que ce serait défavorable. Donc, je vais mettre au voie ces amendements successivement, qui sont les plus identiques, tout à la fois un seul vote avec un avis défavorable de la Commission et un avis de sagesse de la part du gouvernement. Qui est pour ces amendements ? Qui est contre ? Et qui s'abstient ? Ils ne sont pas adoptés. Je mets maintenant en voie l'article unique qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. L'article unique est adopté. Après l'article unique, nous avons un amendement numéro 3, madame Bonnefoy. Nous regrettons en effet que cette proposition de loi pose le principe général d'une dérogation sans contrepartie réelle pour les sports mécaniques et sans aucune disposition permettant d'accompagner notamment les collectivités dans la mise en place de futurs aménagements. Ce texte met ainsi sur un même plan la pratique des activités mécaniques sportives et la protection du voisinage et de la santé humaine. En d'autres termes, la question économique et sportive devra s'apprécier au même titre que celle de la santé des Nuisances au Nord. En renvoyant à un décret le soin de fixer le cadre de ces nouvelles règles, elle prive le législateur que nous sommes de la possibilité de veiller à trouver un équilibre qui satisfasse toutes les parties prenantes. En conséquence, nous estimons donc nécessaire d'introduire une sorte de clause de revoyure. Je précise que nous avons bien conscience que le Sénat tente de limiter au maximum le nombre de rapports. Toutefois, nous considérons que certains rapports sont nécessaires et celui-ci présente un intérêt important qui sera certainement apprécié et attendu par de nombreux riverains de circuits automobiles. Donc je vous engage à voter cet amendement.

faire droit aux demandes de rapport. Donc, la Commission s'oppose à cette demande de rapport. Avis défavorables. Merci, Madame la Ministre. Avis défavorables aussi. Je mets au voie, Monsieur le Président,

si vous me permettez un peu quelque chose de assez traditionnel, n'est pas notre tasse de thé. Et en plus, c'est vrai que les demandes de rapport, ils ne nous sont pas souvent fournies par le gouvernement. C'est vrai qu'on peut les demander mais on n'est pas assuré de les avoir. Et puis deuxièmement sur le suivi. Chaque année il y a une réunion qui se fait pour effectivement suivre l'application des lois et réunion à laquelle j'assiste en tant que président de la commission d'aménagement du territoire et je serai effectivement très très vigilant parce que l'amendement et la réflexion déposée par Nicole Bonnefoy est à mon sens pertinent parce qu'il faut quand même qu'on puisse voir si ce sera bien appliqué ou pas en matière de bruit. Merci. Merci. Je vais donc mettre au voie l'amendement numéro 3 concernant l'article additionnel après l'article unique avec un double AVD favorable de la Commission et du gouvernement qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il n'est pas adopté. J'ai ensuite plusieurs amendements. sur l'intitulé de la proposition de loi et qui font l'objet, ces amendements-là, d'une discussion commune. Le premier amendement, Madame Bonnefoy, numéro 4. actuel de la présente proposition de loi ne semble pas en lien avec le dispositif qu'elle propose. Pire, nous avons le sentiment que ce titre vise à dissimuler quelque peu la vraie nature de ce texte en ne faisant référence à aucun moment au sport mécanique. Nous proposons donc de renommer cette proposition de loi comme suit, proposition de loi visant à instaurer un régime dérogatoire applicable au sport mécanique en matière de prévention des risques liés au bruit. Merci madame la sénatrice, avis de la commission. attendez, pardon, il y a un deuxième amendement en discussion commune. Oui, monsieur Fernic, veuillez m'excuser. Pas de Pas de souci, monsieur le Président. Donc, effectivement, il ne s'agit pas par cet amendement de savoir si on est pour ou contre la proposition de loi, mais simplement de rectifier une erreur de rédaction. pour laquelle je pense que nous allons trouver une rectification consensuelle. Les auteurs de la proposition de loi nous disent qu'à ce jour, je les cite, les circuits de sport mécanique se trouvent soumis à des règles disproportionnées, voire parfois inapplicables, mettant en péril l'avenir des sports mécaniques en France. L'intitulé, vous pouvez le lire à l'écran ici, de la proposition de loi ne reflète donc pas l'objectif poursuivi, or il convient d'être précis sur l'intitulé des textes qui sont soumis au vote du Parlement. Le présent amendement vise à remettre en cohérence l'intitulé et l'objet de la proposition de loi de façon claire et précise. Donc vous avez deux propositions, on pourra choisir la rectification qui est la bonne. Il s'agit bien en notre sens d'une proposition de loi visant à court-circuiter la prévention des risques liés au bruit pour les sports mécaniques, Puisqu'on a tout à l'heure cité Jean Jaurès dont j'ignorais la j'ignorais la passion pour les voitures de course, je répondrai en citant Albert Camus, mal nommé les choses, c'est ajouté au malheur du monde. Je vous remercie pour ces citations. Alors l'avis de la commission par monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, alors l'ajout de l'expression régime dérogatoire dans l'individu et de la proposition n'apparaît pas approprié. Pourquoi ? Parce qu'il n'excupe pas par exception les sports mécaniques de la prévention des risques liés. Au contraire, il aménage la prévention des risques liés au bruit pour rendre pleinement applicable aux sports mécaniques. Dans cet avis défavorable. Pour l'amendement numéro 6, pour les mêmes raisons, l'objet de l'expression « co-circuitiers » n'apparaît pas non plus approprié. Dans cet avis défavorable. Je vous remercie. Avis du Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Sagesse. Décidément, vous faites preuve de beaucoup de sagesse. Je vais mettre aux voix ces amendements avec un avis défavorable de la Commission et un avis de sagesse du gouvernement, qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient Sur l'amendement numéro 6, qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vais maintenant mettre en voie la proposition de loi visant à aménager la prévention des risques liés au bruit. Madame Delattre veut s'exprimer. pas l'occasion de pouvoir parler après le vote. Je voulais remercier encore une fois le rapporteur et son administrateur pour le travail qui a été effectué, remercier l'ensemble des groupes qui soutiennent cette proposition de loi, mais également les groupes qui ne soutiennent pas parce que vous avez pu vous exprimer, nous avons pu échanger et je voudrais vous remercier de l'intérêt que vous avez porté aussi à cette proposition de loi et compte tenu des annonces de vote, je me félicite que cette proposition de loi soit adoptée ou sur le point de l'être par le Sénat et je fais confiance effectivement à la navette pour faire en sorte que ce texte remplisse les attentes de chacune et chacun d'entre nous. Merci. Madame, bonne fois à souhaiter prendre la parole. n'aient pas été retenus pour tout parti. J'ai bien entendu le Président de notre commission de l'aménagement du territoire développement durable sur la l'intérêt qui portait à avoir l'application de la loi. Donc c'est une bonne chose, c'est important. Donc je lui rappellerai au cas où cette analyse de l'application ne se fasse pas parce que la question du bruit est une question majeure. Donc pour l'essentiel de mon groupe, nous voterons contre cette proposition de loi, sachant que quelques-uns dans notre groupe voteront pour la proposition de loi. Monsieur le Président, après le vote, d'accord, je vais mettre au voie l'ensemble de cette proposition de loi qui est pour qui est contre, qui s'abstient, est adopté. Monsieur le Président. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Moi, tout d'abord, je voudrais remercier l'auteur de cette proposition de loi. Merci et remercier le rapporteur. Et vous remercier toutes et tous, parce que pour celles et ceux qui ont voté pour et même celles et ceux qui ont voté contre, Je crois que c'était un débat très intéressant qui permet effectivement de s'exprimer parce que l'histoire du bruit, ce n'est pas quelque chose qui ne doit pas nous interpeller. Effectivement, on doit à ce sujet être particulièrement vigilants. Simplement, je connais Nicole Bonnefoy qui, je sais, ne lâchera rien et je m'engage effectivement et au près de Jacques Fernic aussi à avoir un suivi de ce texte pour effectivement parce qu'en tant que président de la commission d'aménagement du territoire et du développement durable il est aussi important que je puisse avoir une oreille attentive si j'ose m'exprimer ainsi sur les effets néfastes du bruit. Je vous remercie toutes et tous pour votre présence. Merci aussi au service pour le travail effectué parce que cette proposition de loi, on a commencé à l'examiner il y a quelques semaines à peine et puis elle est déjà devant nous et j'espère que l'Assemblée nationale, elle sera suivie correctement pour que l'on puisse la mettre en œuvre. Merci vous toutes pour votre présence et votre attention à cette proposition de loi. Merci. loi. Merci. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre. Monsieur le Président, d'abord une première remarque introductive qui va vous faire plaisir. Lorsque j'ai exprimé mon dernier avis de sagesse, je n'avais pas dissocié l'article 6 pour lequel mon avis était défavorable. Cette précision est en fait, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, je voulais vous remercier de ce temps d'échange, féliciter évidemment Nathalie Delattre pour sa volonté d'essayer de trouver les meilleurs équilibres possibles et d'avoir travaillé avec l'ensemble des services du Sénat auquel je veux également rendre hommage sur un texte et vous dire avec beaucoup de simplicité que Je suis heureuse que le débat puisse maintenant se poursuivre, s'approfondir dans le cadre de la navette parlementaire. On a besoin sur ces enjeux, il s'agit d'un côté de préserver les sports mécaniques, de l'autre de ne rien lâcher sur le terrain de la préservation de la santé publique et de la défense de l'environnement. Et nous avons besoin du législateur, nous avons besoin de la loi pour avancer. Le groupe de travail a montré sa portée. ces limites. Vous l'avez évoqué à plusieurs reprises. Nous voyons aujourd'hui que pour poser les curseurs aux bons endroits, c'est du niveau de la loi dont nous avons besoin. Un grand merci à vous. Merci, madame la ministre. Je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 14h30 pour l'examen du projet de loi de finances pour 2024. La séance est suspendue.